aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles.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 l'examen de la proposition de résolution tendant à mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à simplifier certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux équipements sportifs présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par MM. Dominique de Legge, Christian Manable,

du Sénat sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Il y a du travail ! Elle fait également suite à la mission d'information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales présidée par notre collègue Michel Savin en 2014. Savin en 2014. Quelle est la situation aujourd'hui ? Selon l'Association nationale des élus en charge du sport, l'ANDES, les collectivités territoriales sont aujourd'hui les premiers financeurs du sport, puisqu'elles assurent un peu plus de 12 milliards d'euros de dépenses par an, soit 70 % des financements publics.

conteste les règles en matière de sécurité ou d'accessibilité, la multiplication, l'empilement, et l'application sans discernement de ces règles deviennent aujourd'hui insupportables, leur addition créant

série de normes, à commencer par les normes générales, celles qui s'appliquent aux établissements recevant du public. L'élu local doit ensuite faire face aux normes réglementaires des fédérations sportives. Si l'on peut comprendre que ces dernières ont peu de marge s'agissant d'instructions d'ordre international, on peut en revanche être un peu plus critique lorsque ces recommandations sont dictées par des impératifs commerciaux. Je pense notamment à la « contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public », aux « dispositifs liés à la retransmission télévisée des compétitions », ou aux panneaux publicitaires.

du sport en général. Ces normes soulèvent une difficulté : si elles sont dites « volontaires », les juges les reconnaissent de plus en plus comme des obligations entraînant la responsabilité des gestionnaires en cas de difficultés. Il n'y a donc pas un producteur unique de normes, mais, à un moment donné, au bout de la chaîne, il y a bel et bien un réceptacle unique : les élus locaux. Mes collègues Michel Savin et Christian Manable développeront plusieurs points et pistes d'évolution. Pour ma part, je souhaite insister sur trois points. nous devons passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Trop souvent, la norme est perçue comme une assurance pour se prémunir d'une action en responsabilité en cas d'accident, la réalité de l'usage des équipements et des publics qui les fréquentent étant reléguée au second plan. Deuxièmement, les équipements sportifs sont composés de plusieurs parties, qui répondent à des fonctionnalités particulières et différentes. L'application de la norme doit se faire en tenant compte des usages réels de chacune de ces parties. toute activité humaine étant génératrice de risques, tout doit être fait pour les prévenir. La conception des équipements y contribue bien évidemment. Mais les comportements des usagers doivent être compatibles avec la finalité desdits équipements. De ce point de vue, les responsabilités doivent être mieux partagées, au risque de dissuader les acteurs locaux d'investir. Mes collègues et moi-même avons souhaité adopter une approche pragmatique, en formulant des souhaits dont la réalisation dépendra d'un travail commun de l'administration,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l'a rappelé notre collègue Dominique de Legge, cette proposition de résolution est le fruit d'un travail commun. C'est exact, nous avons tous à coeur de desserrer les contraintes et d'alléger les coûts qui pèsent sur les collectivités territoriales. Les élus locaux le réclament régulièrement et nous devons les entendre. Nous le savons tous, les collectivités territoriales investissent chaque année près de 12 milliards d'euros au bénéfice des 36 millions de pratiquants de notre pays. Ces coûts induits sont surtout le résultat du dynamisme sportif des clubs, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Toutefois, les élus locaux ne comprennent pas toujours d'être sollicités pour investir dans des équipements qui ne sont plus aux normes en raison de nouvelles règles édictées par les fédérations sportives suite du passage d'un club ou d'une équipe d'une division à une autre, ce qui modifie le niveau d'homologation des équipements et impose des investissements importants pour appliquer les normes correspondantes. Comme mon collègue Dominique de Legge, je pense que les élus locaux ne veulent pas forcément moins de normes, mais moins de normes inutiles ; ils veulent la bonne norme au bon endroit. Depuis mars 2009, nous disposons d'une instance de concertation reconnue, légitime, efficace et, surtout, plébiscitée par tous les acteurs, à savoir la Commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, la CERFRES, qui réunit l'État, les collectivités territoriales et le mouvement sportif. On ne peut plus dire que les normes sont « hors-sol » ou édictées au mépris de toute consultation des élus locaux. Nous devons, je le dis devant Mme la ministre des sports, préserver cette instance de dialogue, tout en souhaitant la consolidation de ses prérogatives. Il nous paraît surtout indispensable de changer l'approche entretenue à l'égard des normes, pour qu'elles s'adaptent mieux aux situations concrètes. Selon nous, les normes doivent répondre à deux exigences. Il s'agit tout d'abord d'une exigence de bon équilibre selon les équipements. Nous devons prévoir des normes qui soient fonction de l'usage réel d'un équipement. Cette exigence de bon équilibre des prescriptions s'appliquerait aussi selon qu'il s'agit de manifestations sportives locales, régionales ou nationales, de sport amateur et/ou professionnel. Les normes doivent ensuite répondre à une exigence d'adaptabilité aux situations. On ne peut pas vouloir limiter les coûts sans envisager une utilisation pluridisciplinaire des équipements sportifs. Nous invitons donc les fédérations à dialoguer davantage pour assurer la polyvalence et le partage de leurs équipements. Elles pourraient par exemple s'entendre sur des « guides d'utilisation communs » des salles et des équipements sportifs. L'adaptation des normes commande ensuite à leur application. Les textes des fédérations sportives devraient se borner à fixer des objectifs à atteindre, à charge pour les collectivités territoriales d'en définir les modalités d'application pour y parvenir selon les réalités et les besoins locaux. Elle commande enfin de prévoir une application différenciée des normes et règles d'homologation, selon les différents espaces d'une même infrastructure sportive, pour tenir compte de son usage réel. Je conclurai cette présentation en soulignant que nous-mêmes, en tant que législateurs, devons être pleinement conscients des efforts de simplification que nous exigeons des autres producteurs de normes. La parole

Je rappellerai d'abord que cette proposition de résolution est le résultat de plusieurs mois de travail. Nous avons auditionné tous les acteurs concernés : les grandes fédérations sportives, bien sûr, les ligues professionnelles, les représentants des collectivités territoriales, l'administration des sports, les instances nationales spécialisées, et même les fabricants et équipementiers de l'industrie du sport. Comme mes collègues viennent de le souligner, nous avons souhaité répondre à une demande forte et récurrente des élus des territoires, à savoir la simplification des normes sportives applicables aux collectivités territoriales. C'est précisément l'objet de cette proposition de résolution. La matière étant essentiellement réglementaire, l'instrument de la résolution s'est effectivement imposé comme étant le plus adapté à nos propositions. Dominique de Legge ayant rappelé la philosophie générale du texte et Michel Savin ayant présenté les deux exigences piliers de cette proposition, à savoir la proportionnalité et l'adaptabilité des normes, je me concentrerai sur les points plus techniques. Depuis le 27 mars 2009, une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, la CERFRES, tente d'exercer, avec d'autres élus - les représentants de l'Association nationale des élus en charge du sport, l'ANDES, des départements et des régions des régions - un contrôle sur la production normative des fédérations sportives. Formation restreinte du Centre national pour le développement du sport, le CNDS, la CERFRES est ainsi consultée sur tous les projets de norme nouvelle d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions. Si sa création a permis de circonscrire le champ de compétence des fédérations sportives, de responsabiliser celles-ci et de favoriser la concertation avec les collectivités territoriales maîtres d'ouvrage, des améliorations peuvent encore être envisagées. C'est dans ce cadre, madame la ministre, que nous souhaiterions faire plusieurs propositions, il convient d'allonger les délais d'examen des projets de règlements fédéraux de deux à trois mois, pour donner plus de temps aux différents acteurs. Il s'agit en particulier de permettre, aux fédérations, une « fertilisation croisée » des initiatives et, aux collectivités territoriales, une meilleure évaluation des impacts financiers des normes nouvelles. Deuxième proposition, il nous paraît également important de sensibiliser les fédérations sportives à la nécessité de bien veiller à laisser aux collectivités territoriales un délai raisonnable pour la mise en conformité aux normes nouvelles de leurs équipements ou infrastructures. Il serait par exemple utile que les fédérations élaborent des échéanciers prévoyant une date butoir d'opposabilité des normes nouvelles, qui tiennent compte de la taille de la collectivité, des contraintes locales et des réalités territoriales. En somme, plus de progressivité et plus d'adaptabilité. Troisième proposition, nous souhaiterons envisager, avec les associations d'élus concernées - AMF, AdF, Régions de France, notamment -, un élargissement de la composition de la CERFRES, afin de mieux prendre en compte le monde rural et les intercommunalités, de plus en plus nombreuses

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le rôle et l'importance des collectivités territoriales dans le financement et le développement de la pratique sportive ne sont plus à prouver, les orateurs qui m'ont précédé l'ont très bien expliqué. Et les chiffres sont éloquents Le rôle dévolu aux collectivités pèse d'ailleurs tout particulièrement sur les communes, ce qui rappelle leur position privilégiée de proximité, notamment dans le cadre de l'activité sociale qu'est le sport.

s'il continue à faire des économies sur le dos des collectivités et sur celui des associations, y compris des associations sportives. Cela est d'autant plus inquiétant que le sport amateur souffre bien plus que le sport professionnel, lequel bénéficie également de fonds publics. La loi Bailly adoptée l'an dernier, et dont il faudra dresser un bilan précis, a tenté d'encadrer un certain nombre de pratiques. Le diptyque « mutualisation des dépenses-privatisation des profits » a tourné à plein régime les partenariats public-privé, ces PPP mis en place pour faire sortir de terre ... de véritables gouffres financiers pour les collectivités territoriales Permettez-moi de citer l'Allianz Riviera, à Nice, ou la MMArena, au Mans. Et même un stade comme le Groupama Stadium, à Lyon, a fait l'objet, au titre des infrastructures, d'un investissement public de 200 millions d'euros, dont les retombées pour la communauté nationale sont encore à prouver, d'autant que les sommes engagées pourraient être plus utiles dans d'autres chantiers à vocation sportive. Je pense tout particulièrement au sport amateur, exsangue aujourd'hui, car mis à mal de la non-compensation de la suppression de la réserve parlementaire, dont 10 millions d'euros allaient aux associations sportives ! L'importance des collectivités territoriales dans le dynamisme de la pratique sportive en France, avec toutes les vertus sociales, civiques, émancipatrices et économiques que cela comporte,

effet, les fédérations sportives nationales et internationales sont toujours décisionnaires, dans l'élaboration des normes. Je le rappelle, ces dernières ont connu une inflation importante, avec 400 000 normes sportives, dont seulement un peu plus de 8 % sont des normes dites « AFNOR

impliquera des coûts supplémentaires pour les communes concernées dans le cadre de l'organisation des matchs mais aussi de la maintenance des stades et des pelouses. Venons-en au fond de la proposition de résolution. Comme je le disais à l'instant, le renforcement des rôles de la CERFRES recueille totalement notre assentiment. À ce titre, la question des « normes grises » devra faire l'objet d'un examen attentif. Je suis toutefois un peu dubitatif sur le principe d'une participation financière des fédérations aux travaux de mise aux normes des équipements. En réalité, ce n'est pas le principe qui me pose problème, mais les conditions de sa mise en application. Ma première interrogation concerne le rôle des ligues professionnelles dans le processus. Il ne s'agirait pas que les fédérations sportives se retrouvent à supporter le poids financier de normes édictées pour les ligues. Pour ne prendre qu'un exemple, ce sont ces dernières qui négocient les droits télévisés et font appliquer des normes à finalité commerciale et économique aux équipements, pour permettre la captation audio et vidéo des rencontres. Il s'agit d'un vrai questionnement. Mon autre interrogation porte sur les mécanismes qu'une transcription législative de la résolution pourrait mettre en place, notamment pour s'assurer que le sport professionnel ne capte pas l'essentiel de la contribution financière des fédérations pour la normalisation des équipements.

En effet, si je ne doute pas que certaines normes sont inadaptées et malvenues, je m'interroge sur la question des équipements, ou plutôt la nature de ces derniers. Nos collègues le savent, les collectivités ont déjà lancé depuis plusieurs années des mutualisations

Cela permet justement de faire sortir de terre puis d'entretenir des équipements massifs, qu'une collectivité seule ne pourrait financer et « remplir » avec ses seuls administrés. Toutefois, je pense qu'il y a un point d'équilibre à trouver, surtout s'agissant des petits équipements, pour que chaque commune dispose des infrastructures nécessaires pour ses habitants, mais aussi pour ses écoles. Concrètement, il ne faut pas que cette mutualisation conduise à une nouvelle raréfaction des équipements,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je partirai d'un constat simple : trop de normes en matière sportive étouffent les élus locaux que nous avons été et que nous sommes encore, et deviennent la hantise des collectivités. Toutefois, la situation évolue et le travail visant à les rationaliser s'inscrit directement dans l'action, plus globale, de « chasse aux normes » appliquées aux collectivités territoriales que mène le Sénat, « lanceur d'alerte » en ce domaine depuis la XIII législature. Il convient de saluer l'importante réflexion menée par plusieurs de nos collègues sur le sujet, dans un contexte d'érosion tendancielle des dotations versées par l'État aux collectivités. Le débat perdure et, pour revenir au sujet qui nous intéresse, les normes sportives, j'insisterai sur la qualité de l'ensemble des travaux, souvent menés en concertation au sein de notre Haute Assemblée. Au-delà de l'image réductrice de « dépoussiérage » d'un corpus législatif et réglementaire pléthorique, résultat de la sédimentation d'une longue histoire juridique et d'une accumulation de textes foisonnants produits par de par de trop nombreux organismes, l'inflation normative et ses conséquences financières renvoient à une évolution sociétale induisant de nombreux facteurs de régulation. C'est ainsi qu'en matière de pratiques et d'équipements sportifs les différents régimes juridiques mêlent normalisation, de type AFNOR, CEN ou ISO, et réglementation obligeant les collectivités à mettre en conformité les équipements avec les normes édictées par les fédérations sportives, qu'il s'agisse des dimensions du terrain, de l'éclairage, des vestiaires, des tribunes et que sais-je encore. Je souhaite m'attarder

être un outil de l'efficience législative et du choc de simplification. Leur mode d'élaboration collectif leur confère un statut de règle de l'art tout à fait pertinent que nous nous devons d'exploiter, sans nous départir bien évidemment d'une certaine objectivité, dans la mesure où elles ne sont pas sans importance sur les obligations des collectivités. Cet ajustement fait, l'action en faveur du contrôle des normes obligatoires relatives aux équipements sportifs des collectivités territoriales s'est améliorée, mais reste encore insuffisante. Ce contrôle est aujourd'hui devenu essentiel, car il n'est plus à démontrer l'impact négatif que le foisonnement normatif fait peser sur les collectivités en termes financiers, logistiques, voire en termes de responsabilité. Quels sont les avantages à baisser les normes en matière de sport ? L'avantage est d'abord logistique. Il devient ainsi nécessaire de clarifier et d'harmoniser l'enchevêtrement de normes complexes produites par des organismes trop nombreux et souvent peu coordonnés.

les normes réglementaires, produites, elles, par les fédérations sportives délégataires incluant exigence de pratiques sportives et recommandations d'ordre commercial non obligatoires, et les normes d'homologation. Il est urgent de procéder à une rationalisation des normes, afin que celles-ci soient non plus additionnelles mais complémentaires et cessent de peser aussi lourdement sur le budget des collectivités territoriales.

et les plus grandes pourvoyeuses d'équipements sportifs. Or, eu égard au contexte budgétaire plus que contraint que nous connaissons aujourd'hui, nous ne pouvons faire l'économie d'un travail méticuleux de réduction des normes. À ce titre, les projections de l'ANDES sont édifiantes

occulter la question fondamentale du bien-fondé des règles de sécurité. J'en viens maintenant aux nécessaires améliorations à apporter dans ce domaine aux fins de pragmatisme et de rationalisation.

faire légitimement entendre leur voix pour l'élaboration des réglementations édictées par les fédérations sportives. Il faut cependant aller plus loin : des progrès restent à faire. Je n'énumérerai pas l'ensemble des propositions du texte en termes d'adaptabilité et de proportionnalité, mais j'insisterai sur certains points. en premier lieu, de renforcer la légitimité ainsi que l'importance de la CERFRES auprès des fédérations sportives, en rendant ses avis obligatoires et non plus consultatifs. lui laisser le temps nécessaire pour examiner les projets de règlement qui lui sont soumis et mener une analyse pertinente. Il serait par ailleurs souhaitable que la CERFRES puisse être saisie de l'examen des projets des ligues professionnelles, qu'un système d'évaluation des normes soit mis en place et que, plus généralement, l'ensemble des dispositions des fédérations et ligues présentant des conséquences financières et logistiques importantes pour les collectivités soient examinées par la commission. Enfin, un constat s'impose : la CERFRES a très peu saisi le CNEN, le Conseil national d'évaluation des normes, pour faire entendre sa décision à une fédération qui irait à l'encontre de son avis. Faisons-en sorte qu'une telle possibilité devienne un réflexe.

Enfin, je tiens à remercier et à féliciter les auteurs de cette proposition de résolution, nos collègues Dominique de Legge, Michel Savin et Christian Manable, pour l'excellent travail réalisé. La parole

proposition de résolution, j'en reviens à la quatrième. Il nous paraît indispensable de réfléchir à la création de groupes de travail qui associeraient en amont la CERFRES et les fabricants d'équipements sportifs, afin de bénéficier de leur expertise. C'est d'ailleurs, je dois le dire, une demande forte de la part car ils sont prêts à jouer le jeu de la mutualisation et de la polyvalence des équipements sportifs. Cinquième proposition : selon nous, la CERFRES devrait pouvoir se saisir des « normes grises

Septième proposition : ses compétences d'évaluation mériteraient d'être consolidées, par exemple la mise en place d'une révision régulière des normes tenant compte de l'expérience des collectivités territoriales.

Cette faculté est aujourd'hui largement inutilisée, alors même que le CNEN plaide pour une meilleure articulation et un échange plus régulier entre ces instances. Neuvième proposition, enfin : nous voudrions inciter la CERFRES à s'autosaisir, à la demande d'une collectivité territoriale, d'un problème rencontré concernant une norme fédérale.

Premier péché capital : les coûts élevés. Les coûts des équipements exigés par les fédérations et les ligues vont de plusieurs dizaines de millions d'euros, pour les stades de football de Ligue 1, à des sommes certes plus modestes, mais qui impactent néanmoins les budgets locaux.

quatre portes de piste n'étaient pas suffisantes. Deux portes ont ainsi dû être ajoutées à Lille Métropole, en remplacement de panneaux de rambarde, pour un coût de 3 000 euros hors taxe. Deuxième péché capital : l'instabilité normative. Les fédérations ne cessent de perfectionner leurs normes, les modifiant sans s'interroger sur les conséquences de ces modifications sur les équipements existants.

La mise aux normes entraîne un coût compris entre 2 000 et 10 000 euros suivant les équipements- parquet, sol souple, etc. -et n'apporte pas la preuve d'une légitimité indéniable : il n'y a toujours pas d'uniformité mondiale- les tracés diffèrent selon les ligues et selon les pays. Cela signifie-t-il qu'un nouveau changement sera obligatoire dans le futur ? Troisième péché capital : l'« aristocratie » normative. Dans le monde des fédérations, l'aristocratie ne se manifeste pas par l'affichage de quartiers de noblesse, mais par la qualité des locaux d'accueil, qui varie selon les niveaux de jeu. Il en est ainsi de la taille des vestiaires réservés aux arbitres, qui augmente en fonction du classement sportif. Malgré un investissement de 1 million d'euros pour la réalisation d'un terrain de football en revêtement synthétique dans son complexe sportif Maurice-Fouque, la ville de Caen voit ce même terrain déclassé par la Fédération française de football de la catégorie 4 à la catégorie 5, en raison de la dimension des vestiaires des arbitres. Si la ville n'avait pas réalisé de travaux sur l'aire de jeu et l'éclairage, le terrain serait resté en catégorie

pour les compétitions de niveau « championnat de France », il est nécessaire de disposer d'un local antidopage, de quatre vestiaires et de deux vestiaires « arbitres »- 1 500 euros d'amende par match sont prévus si la salle n'est pas conforme.

ces zones doivent être plus ou moins éclairées suivant le classement de l'équipement. Cette réglementation engendre une augmentation de la puissance électrique exigée. Le dispositif technique est difficile à installer lorsque la structure de base ne comporte pas de mâts assez grands ou le câblage nécessaire ; en cas d'accession à une compétition nationale, aucune dérogation ne peut pourtant être accordée. Dans ce cas, le club doit chercher un nouveau stade. péchés capitaux, j'en viens aux incompatibilités normatives. L'absence de toute forme d'harmonisation entre les normes émises par les différentes fédérations rend très difficile l'usage polyvalent d'un même équipement. Ainsi, le basket-ball, le handball et le volley-ball ont des exigences différentes et souvent incompatibles, mais le summum du ridicule, nous l'avons rencontré, lors de notre enquête, lorsque, dans une même salle où l'on pratique le badminton,

Des normes sportives peuvent ainsi aller à l'encontre des dispositions de la loi Handicap ou de la loi Grenelle II. Le code du sport impose une pente des sols de 3 % à 5 % pour éviter les stagnations d'eau,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec plus de 250 000 équipements sur leurs territoires, les collectivités locales sont les premiers propriétaires d'espaces dédiés au sport. elles sont soumises à l'application de plus de 400 000 normes, réglementations et prescriptions, relatives aux capacités d'accueil des équipements, à la forme des chaises d'arbitre, dont vous parliez à l'instant, à la disposition des terrains, au confort des installations, à l'éclairage et à beaucoup d'autres choses- je ne saurais épuiser cette liste, qui est presque une litanie. L'application d'un tel stock normatif, en constante augmentation, n'est pas sans conséquence sur les finances locales, d'autant plus que ces normes réglementaires s'appliquent aussi bien aux plus petites communes rurales qu'aux grandes métropoles. L'Association nationale des élus en charge du sport a chiffré le coût induit par ces normes à 6 milliards d'euros pour les collectivités entre 2008 et 2014. Selon l'OCDE, le fardeau normatif de la France, tous secteurs confondus, s'élève à 60 milliards d'euros par an. La simplification normative est donc, entre autres, un enjeu de compétitivité pour les territoires. Dans un contexte de raréfaction des ressources budgétaires, cette proposition de résolution représente une libération réglementaire et budgétaire pour les élus locaux.

La lutte contre l'inflation normative est une nécessité de longue date. Le stock du droit national applicable en France a augmenté de 50 % en vingt ans. Or, comme le disait Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires »- cette formule me paraît s'appliquer aussi aux normes réglementaires. Face à des contraintes de plus en plus nombreuses, nous appelons de nos voeux une révolution réglementaire. Il faut absolument privilégier la qualité, la souplesse et l'adaptabilité du droit à l'amoncellement de normes inapplicables ou inutiles. C'est là, au sein de l'État de droit qui est le nôtre, une condition indispensable pour bâtir la nouvelle société de confiance, laquelle reposera, comme cette proposition de résolution, sur les principes de responsabilité, de concertation et de subsidiarité.

le texte qui est soumis ce jour à l'approbation de notre Haute Assemblée résulte du travail conjoint de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et de la commission de la culture. Il illustre bien la façon dont le Sénat peut oeuvrer, au service de nos territoires, dépassant les clivages partisans. Le Sénat s'est saisi du champ de la simplification des normes applicables aux collectivités, remplissant ainsi la fonction que lui assigne le quatrième alinéa de l'article 24 de notre Constitution. La présente proposition de résolution porte spécifiquement sur les normes applicables en matière de pratique et d'équipements sportifs. Celles et ceux d'entre nous qui ont été maire ou adjoint aux sports ont immanquablement été confrontés à cet enchevêtrement réglementaire, à son instabilité, à ses paradoxes voire à ses contradictions, qu'il s'agisse des mesures de sécurité, d'accessibilité, de respect de l'environnement ou de l'ensemble des règles encadrant une discipline et ses compétitions.

Ce coût, l'ANDES l'évalue à 6 milliards d'euros sur la période 2008-2014. Comme le souligne l'exposé des motifs, les normes émanent certes de l'exécutif et du législateur, mais sont aussi le fait des fédérations sportives délégataires. Nos anciens collègues Alain Lambert et Jean-Claude Boulard avaient déjà pointé, il y a cinq ans, dans leur premier rapport, « les sept péchés normatifs des fédérations sportives Ils qualifiaient de « dangereuse » la distinction entre le pouvoir normatif des fédérations et l'obligation de payer des collectivités territoriales. Il pourrait donc être légitime de réfléchir à des aménagements de ce pouvoir normatif accordé aux fédérations sportives, portant sur les aires de jeu, mais également sur les espaces dédiés aux sportifs. Aujourd'hui, il est vrai que les collectivités ont peu de prise sur la réglementation applicable à l'immense majorité des 330 000 équipements, espaces et sites dont elles sont pourtant propriétaires. En outre, si le pouvoir réglementaire des fédérations ne concerne concerne pas les demandes d'ordre commercial, il n'est pas rare que les ligues professionnelles édictent des prescriptions qui débordent du cadre prévu par la loi les fameuses « normes grises ». Il faut aussi, à cet égard, souligner le rôle et les demandes des diffuseurs. Il existe enfin une troisième source réglementaire : les normes d'homologation, par exemple celles de l'AFNOR, Sans remettre en cause leur bien-fondé, nous constatons que ces dernières sont souvent considérées par le juge comme des normes impératives, ce qui peut être de nature, en cas d'accident, à engager la responsabilité pénale des élus et des collectivités. Or nous savons- Or nous savons- et la consultation récemment menée par la délégation aux collectivités territoriales sur le statut de l'élu nous le confirme -que la question de la responsabilité des élus est un motif d'inquiétude, voire un frein à l'engagement municipal.

Depuis sa création, en 2009, cette instance collégiale réunissant État, collectivités et mouvement sportif a conduit un travail minutieux contre la surinflation normative. dynamique doit être encouragée et approfondie, en allongeant les délais de consultation, ou en permettant à la CERFRES de s'autosaisir. La composition de la commission pourrait aussi être revue pour mieux prendre en compte le monde rural et les intercommunalités. une meilleure articulation avec les travaux conduits par le CNEN, telle qu'évoquée dans la proposition de résolution, ne pourrait être que bénéfique. La production normative des fédérations sportives doit également évoluer. de résolution développent deux exigences, de proportionnalité et d'adaptabilité, qui sont empreintes de bon sens. Doit-on avoir les mêmes exigences pour un championnat régional et pour une compétition internationale ? Évidemment, non Doit-on encourager le multiusage des équipements par une harmonisation des normes ? À l'évidence, oui. Enfin, le texte- c'est une de ses principales innovations -propose d'associer les fédérations sportives au financement de certaines modifications induites par les changements réglementaires qu'elles imposent, selon le principe du « prescripteur-payeur ». L'aggravation des contraintes qui pèsent sur nos collectivités appelle l'intervention du législateur et de l'exécutif. collègues, le précédent quinquennat avait vu la mise en oeuvre du « choc de simplification », avec des avancées en définitive bien réelles, mais largement insuffisantes. L'actuel gouvernement a lancé son propre plan, comme en témoigne la règle du « deux pour un » ou le programme Action publique 2022. Je relève néanmoins un aveu, fait par Alain Lambert lors de son audition, à la mi-janvier, par la délégation aux collectivités territoriales. Il soulignait une « volonté politique sincère mais redoutait « un sentiment de l'administration centrale considérant que le système ne fonctionne " pas si mal ", et qu'il semble inopportun de changer un système assez équilibré Dans ce contexte, la présente proposition de résolution est donc opportune et utile, car elle se fait l'écho des difficultés rencontrées dans nos villes et dans nos villages. L'ensemble du groupe du RDSE y souscrit pleinement. Nous invitons désormais le Gouvernement à s'emparer de ces travaux pour, à son tour, permettre une évolution des pratiques et de la réglementation en vigueur. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous réunit aujourd'hui est un texte de simplification normative. Depuis quelques années, et davantage encore ces derniers mois, sous l'impulsion du président Gérard Larcher, le Sénat travaille à la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Les élus locaux réclamaient cet élan depuis longtemps simplification des normes dans le domaine de l'urbanisme ou dans celui du service public d'eau potable, entre autres. Mais le domaine que nous traitons aujourd'hui est celui du sport, domaine qui me tient à coeur. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication et la délégation aux collectivités territoriales se sont engagées dans le processus de simplification des normes sportives il y a un an. Elles ont constitué un groupe de travail, et je remercie les rapporteurs de ce groupe, MM. Dominique de Legge, Christian Manable et Michel Savin. Savin. À la suite des tables rondes organisées avec des représentants de fédérations sportives, d'associations d'élus locaux, d'administrations de l'État et d'équipementiers, la proposition de résolution que nous examinons cet après-midi a été élaborée. Elle vise à mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à simplifier certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux équipements sportifs. Nous ne pouvons qu'unanimement approuver ce texte. Comme nous le savons, on ne compte plus les normes, réglementations et prescriptions applicables aux quelque 250 000 équipements, espaces et sites sportifs dont les collectivités territoriales sont propriétaires. Soulignons que les collectivités territoriales sont aujourd'hui les premiers financeurs du sport, assurant 70 % des financements publics, et surtout les premiers propriétaires d'infrastructures sportives en France. Sur le terrain, les normes pleuvent. Les élus locaux sont souvent submergés. Nous devons agir pour faire en sorte de diminuer cette pression normative. La volonté parlementaire de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales est partagée par le Gouvernement. À ce titre, le Premier ministre a demandé à MM. Alain Lambert et Jean-Claude Boulard d'identifier, en coordination avec les ministères, des simplifications du stock de normes applicables aux collectivités. Le programme Action publique 2022 comporte par ailleurs un chantier de simplification. Plusieurs travaux récents recommandent d'agir pour une simplification dans le domaine du sport. Je citerai notamment le rapport de MM. Alain Lambert et Jean-Claude Boulard sur la lutte contre l'inflation normative, remis en mars 2013, le rapport d'avril 2014 de la mission commune d'information du Sénat sur le sport professionnel et les collectivités territoriales, présidée par notre collègue Michel Savin, et un rapport publié en 2015 par l'Inspection générale de l'administration, l'IGA, et l'Inspection générale des affaires sociales, Dans ce domaine du sport, les élus locaux se trouvent constamment face à des normes nouvelles, normes issues des fédérations sportives, du Gouvernement, du Parlement, normes d'homologation du type AFNOR, toutes issues, donc, de producteurs autonomes de normes. Je me félicite de l'existence de la Commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, qui exerce un contrôle sur la production normative des fédérations sportives. Cette commission est à consolider. Il s'agit de l'unique instance de dialogue associant élus et représentants des fédérations sportives. du texte qui nous est soumis proposent de renforcer la composition et les attributions de la CERFRES. L'allongement des délais d'examen des projets de règlements fédéraux me semble également une aide nécessaire aux collectivités. Les fédérations doivent veiller à laisser du temps à ces dernières pour qu'elles Comme cela a été rappelé- c'est un point majeur de ce texte -, la proposition de résolution vise également à encadrer la production normative des fédérations sportives selon des principes de proportionnalité et d'adaptabilité. Je citerai un problème récurrent : les changements de divisions ou de catégories sportives pour les clubs. Lorsqu'une équipe change de division, les normes qui s'appliquent au club deviennent différentes et la collectivité doit alors fournir de nombreux investissements pour s'y conformer, dans des délais contraints. Ces évolutions sont très difficiles à assumer financièrement, en particulier pour les petites collectivités. Pour Pour que la norme sportive réponde à un souci d'adaptabilité, il serait nécessaire que les infrastructures soient multiusage et non réservées à un sport unique. L'exemple du nombre de chaises d'arbitre aussi élevé que le nombre de sports pratiqués dans le gymnase est aberrant. Il arrive même que les normes s'avèrent contradictoires. Les fédérations sportives doivent donc dialoguer, afin d'harmoniser leurs normes. Le futsal a, par exemple, su s'adapter, en reprenant certaines lignes du terrain de handball. L'usage polyvalent d'un même équipement est certes parfois difficile, mais il reste, en la matière, beaucoup d'efforts à faire. Les fédérations sportives sont exigeantes ; nous ne pouvons le leur reprocher. Mais, en raison de leur caractère évolutif, les normes sont instables. Encourageons donc une meilleure adaptabilité. Concernant le nécessaire dialogue entre les fédérations, je souhaite saluer la démarche du Comité international olympique s'agissant de la nouvelle procédure de candidature, applicable aux jeux Olympiques d'hiver de 2026. Cette procédure s'appuie désormais sur un dialogue approfondi entre le CIO, les villes et les comités nationaux olympiques, et prévoit d'importantes réductions budgétaires. Le dialogue porte ses fruits. Il devient urgent de l'encourager, notamment en faveur des collectivités locales. Un mot, enfin, sur l'état des finances de nos collectivités locales. Les normes sportives impactent encore un peu plus ces finances déjà mises à mal- nos collectivités subissent en effet, malheureusement, les politiques successives des gouvernements qui aggravent leur état de santé financière. Une majorité d'entre nous, sur ces travées, dénonce les 13 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités sur cinq ans, l'abandon brutal de 120 000 emplois aidés, la fin annoncée de la taxe d'habitation, qui affectent durement la santé financière des collectivités territoriales et mettent en péril leurs projets locaux. Ce texte va dans le sens d'une aide apportée à nos collectivités ; il constitue un pas supplémentaire dans le processus de simplification. Nous devons poursuivre cette dynamique. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui se situe dans la continuité des travaux engagés par le Sénat pour lutter contre l'inflation des normes. à des propositions de résolution dédiées aux entreprises, à l'urbanisme et à la construction, à l'agriculture, à la gestion de l'eau et à la vie économique, cette proposition de résolution traite des normes liées à la pratique et aux équipements sportifs. Il s'agit, là encore, de simplifier, d'harmoniser, de mutualiser, d'évaluer, de ne garder que le nécessaire et l'utile, dans un esprit de maîtrise des coûts. Nos collectivités territoriales sont en effet impactées au quotidien par le poids de ces règles de toute nature : plus de 400 000 normes pour 250 000 équipements, espaces et sites sportifs dont elles sont propriétaires. L'obscurité, L'obscurité, l'incompatibilité, l'obsolescence des contraintes normatives dans le domaine du sport, ainsi que la pression d'intérêts commerciaux, ont été souvent dénoncées, notamment par le Conseil national d'évaluation des normes,

Mais le tri n'est pas facile, et la tâche est complexe, pour ne garder que la bonne norme, à sa juste place, au moment adéquat. Le Gouvernement, pour sa part, s'y est attelé sans tarder. Dès juillet 2017, le Premier ministre a décidé que, pour toute nouvelle norme, deux seraient supprimées. Dans le cadre d'un programme de transformation de l'action publique, il a confié au président du Conseil national d'évaluation des normes, Alain Lambert, et à notre ancien collègue Jean-Claude Boulard

Le comité de pilotage sur la gouvernance du sport contribue aussi à cette réflexion. Installé par Mme la ministre des sports à l'occasion du dernier congrès des maires et des présidents d'intercommunalité, il réunit les acteurs de la vie sportive pour imaginer un nouveau cadre institutionnel et organisationnel du sport en France. Par ailleurs, depuis le 1 janvier, les préfets de certains départements peuvent, à titre expérimental, déroger pendant deux ans à des normes dans plusieurs domaines, dont le bâtiment et les activités sportives. C'est le cas pour mon département, Mayotte. Cette initiative est particulièrement bienvenue : alors que plus de la moitié de notre population a moins de vingt ans, les équipements sportifs sont quasi inexistants sur notre île. De tels équipements doivent pouvoir être construits rapidement et simplement, être utiles au plus grand nombre et adaptés au climat tropical. Les recommandations proposées à notre vote se veulent pragmatiques et concrètes. Elles visent essentiellement à renforcer le rôle de la Commission d'examen des projets de règlement fédéraux relatifs aux équipements sportifs, la CERFRES. Il s'agit de conforter son rôle central d'instance de concertation entre l'État, les élus et le monde sportif, en améliorant son fonctionnement et en élargissant son champ de compétences. du fonctionnement, les auteurs du texte envisagent d'élargir le collège pour mieux prendre en compte le monde rural et les intercommunalités, d'allonger de deux mois à trois mois les délais d'examen des projets de règlement fédéraux et de réactiver la procédure de saisine du Conseil national d'évaluation des normes, le CNEN. Ils proposent de réfléchir à la création de groupes de travail associant en amont la Commission et les fabricants d'équipements sportifs,

en principe non obligatoires, mais qui ont de fait un impact sur l'exploitation de l'infrastructure. La proposition de résolution vise également à encadrer la production normative des fédérations sportives, selon les principes de proportionnalité, d'adaptabilité et de mutualisation. Elle insiste sur la nécessité de laisser aux collectivités un délai raisonnable pour la mise en conformité des équipements. Soucieux de ne pas altérer le développement de l'offre sportive, tout en préservant les finances locales, les auteurs de la proposition de résolution respectent donc l'esprit de la démarche générale de simplification et

Il est un autre sujet qui mériterait un débat plus approfondi, et sur lequel nous émettons donc des réserves. Je pense à la demande d'ajout d'une nouvelle norme : celle du prescripteur-payeur, qui vise les fédérations. En fait, elle s'applique déjà en partie dans le cadre des conventions de mise à disposition des équipements entre les propriétaires et les utilisateurs. Il nous semble important au préalable d'en circonscrire le champ d'application en l'envisageant notamment pour les « normes grises » et de réfléchir aux modalités de sa mise en oeuvre. Pour ces raisons, le groupe La République En Marche s'abstiendra. C'est bien

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de groupe, Claude Malhuret, pour remercier les auteurs de cette proposition de résolution, Dominique de Legge, Michel Savin et Christian Manable. Ce texte cible plus particulièrement les recommandations édictées par les fédérations et propose de renforcer les prérogatives de contrôle de la Commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Dans un contexte d'inflation normative et de restriction budgétaire, il s'agit en effet de mieux discerner les normes véritablement utiles des contraintes coûteuses et inadaptées aux situations locales, ces « normes grises » produites par les fédérations sportives et dont il convient d'encadrer la prolifération. Cela implique, d'une part, d'encadrer la production normative des fédérations selon un principe de proportionnalité et, d'autre part, d'instaurer une exigence d'adaptabilité des normes, afin d'autoriser une certaine souplesse dans leur application, selon les contraintes locales. Le besoin d'espaces sportifs polyvalents est, par exemple, une demande forte des élus locaux. Enfin, la règle du « prescripteur-payeur » est intéressante dans la mesure où elle inviterait les fédérations à la modération normative et allégerait les charges pesant sur les finances locales. Il s'agit évidemment non pas de ne plus réglementer, mais de mieux réglementer, en évaluant systématiquement l'impact de chaque nouvelle norme à l'aune des bénéfices apportés aux utilisateurs et des charges financières induites. induites. Il est proposé de renforcer la composition et les attributions de la Commission. À ce titre, il me paraît tout à fait pertinent d'étendre sa composition aux intercommunalités et aux associations d'élus ruraux, afin qu'elle reflète davantage les réalités locales de gestion des établissements sportifs. Il s'agirait également de renforcer la portée du contrôle et le pouvoir d'autosaisine de la Commission en étendant son champ d'action aux recommandations non obligatoires, dites « normes grises », et aux décisions relatives aux compétitions sportives susceptibles d'impacter l'exploitation d'un équipement. Ces différents éléments amènent le groupe Les Indépendants à apporter tout son soutien à cette proposition de résolution, qui s'inscrit pleinement dans le projet d'une nouvelle société de confiance. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 24 de notre Constitution dispose que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République Haute Assemblée est donc bien dans son rôle aujourd'hui en soutenant avec force une légitime demande émanant depuis de nombreuses années des élus locaux : la simplification des normes réglementaires applicables aux collectivités territoriales, notamment dans le domaine de la pratique et des équipements sportifs La proposition de résolution consensuelle que nous examinons aujourd'hui a pour origine un questionnaire diffusé en 2014, lors du Congrès des maires. le constat du rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative, rédigé par Alain Lambert et Jean-Claude Boulard, a fait apparaître l'absurdité dans certains cas du mécanisme des dépenses à finalité sportive. Force est de constater que le sujet des normes relatives aux équipements sportifs des collectivités est devenu de plus en plus délicat à gérer pour nombre d'élus locaux. La multiplication de ces normes conduit en effet les collectivités à ne plus pouvoir distinguer les mesures utiles des contraintes coûteuses et sans objet. Par ailleurs, elle impacte lourdement les finances communales ou intercommunales, alors même que nous sommes en pleine période de disette budgétaire. Quel que soit le problème soulevé, on ne se pose pas de question : l'administration opte toujours pour le degré le plus contraignant

! Bien entendu, aucun élu ne remettra en cause les exigences de sécurité et d'accessibilité dans les pratiques sportives. Mais il est aujourd'hui évident que les limites sont dépassées. Il est grand temps de remettre les choses à plat. Ajouter les textes les uns aux autres sans jamais s'interroger sur la cohérence de l'ensemble conduit à des situations kafkaïennes.

C'est même ce qui irrigue cette proposition de résolution, déposée par nos collègues Dominique de Legge, Christian Manable et Michel Savin, proposition à laquelle je m'associe bien volontiers. Je souhaite également rappeler ici quelques préalables incontournables pour aboutir. Il est en effet indispensable que chaque partie au dossier contribue à son propre niveau à la dynamique d'ensemble et cesse de travailler en silo ! Par exemple, les fédérations doivent effectivement dialoguer entre elles. Bon nombre de celles-ci y sont prêtes.

La proposition de résolution le recommande, et c'est une excellente chose. Permettre également la possibilité d'autosaisine de la CERFRES est une bonne idée, sous réserve toutefois que l'ensemble des fédérations sportives lui soumettent leur règlement. Et c'est là que Et c'est là que le bât blesse, car rien ne les y oblige ! Pour mettre fin à la gabegie d'argent public, il n'y a pas d'autre moyen que de responsabiliser, y compris financièrement, les acteurs. La mise à contribution des fédérations et des ligues selon le principe du « prescripteur-payeur » est la mesure qui s'impose. Imputer pour moitié tout surcoût financier aux fédérations sportives qui en seraient à l'origine les inciterait sans aucun doute à la modération. Cette mesure est déjà en place depuis plusieurs années à la Fédération française de football, le fonds d'aide au football amateur, le FAFA, qui aide la création ou la mise en conformité d'installations sportives. Elle produit de bons résultats. Généralisons-la ! L'adaptabilité, la mutualisation et la proportionnalité recommandées dans cette proposition de résolution sont des critères incontournables. Aussi, madame la ministre, je suis certain que vous aurez à coeur de vous attaquer avec pragmatisme à une situation qui pénalise nos collectivités et nuit au développement de la pratique sportive. Faire un état des lieux exhaustif des textes actuels pour détecter les incohérences, les doublons et les mesures inutiles est la première des priorités responsabiliser financièrement les acteurs, la seconde. On agirait ainsi sur le stock et sur le flux, ce qui, chacun d'entre nous le sait, est la seule méthode valable lorsque l'on veut simplifier les règles en vigueur. La parole est

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne suis pas cosignataire de cette proposition de résolution. Pourtant, au regard de son contenu, j'aurais évidemment pu la soutenir dès le début ; je ne manquerai d'ailleurs pas de le faire dans quelques minutes, en l'adoptant. En effet, sans être une spécialiste du sport, je suis, comme une grande partie d'entre vous, une élue locale qui assiste à de très nombreuses manifestations sportives. Je dirais même que le sport est devenu, dans les territoires ruraux, comme dans les communes plus importantes, notamment celles contenant des zones urbaines sensibles, un élément fédérateur qui rassemble la population sans distinction. Le sport crée un creuset social indispensable à la vie et au développement de tous les territoires de la République. Pour ce faire, les élus locaux, au premier rang desquels les maires, sont des moteurs. La création d'un espace sportif, comme un stade de football ou un terrain de pétanque, est un des moments forts de la concrétisation de la vie municipale ou intercommunale.

Cette addition d'obligations, ce millefeuille de normes, a pour conséquence d'alourdir le coût et l'entretien de ces équipements, d'autant plus que l'argent de l'État, le Centre national du sport, se raréfie sensiblement. L'État, la région et, de plus en plus souvent, le département consacrent leurs aides aux projets dits « structurants », mais pas forcément au fonctionnement. Bref, nous, élus locaux, sommes coincés par une équation de plus en plus insoluble avec, d'un côté, le renforcement des coûts et, de l'autre, la baisse des aides, notamment de l'État. Demain, avec la baisse des dotations et le renforcement des normes, seuls quelques équipements régionaux pourront prétendre à accueillir des compétitions sportives et à être éligibles aux aides publiques. Je ne peux pas accepter cette vision d'une centralisation sportive. Bien entendu, nous devons faire respecter des normes, et en premier lieu les normes sécuritaires, notamment face aux potentielles attaques terroristes, comme notre pays en a malheureusement connu ces derniers jours, mais aussi aux débordements de certains publics.

La commune ou l'EPCI, maître d'ouvrage et principal financeur du projet, doit pouvoir, avec le comité ou la ligue de la fédération compétente, trouver des moyens d'éviter les coûts inutiles. Comment accepter des normes de confort alors que nos collectivités ont parfois du mal à mobiliser de l'agent public pour l'aide sociale d'urgence ? En effet, comment envisager que les normes lumineuses, par exemple, soient les mêmes à Brest ou à Tourcoing que dans le sud de la France, où l'ensoleillement est plus important, et nier parallèlement les exigences environnementales en matière d'éclairage nocturne Il serait d'ailleurs nécessaire de mettre en adéquation ces normes avec les normes environnementales, comme cela avait d'ailleurs été évoqué dans le cadre de la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, qui avait été adoptée en 2011 sous la présidence de M. Sarkozy.

capacités d'accueil du public plus nombreux, sans compter les exigences des fédérations et des médias. Ainsi, comme le préconise la proposition de résolution, il faut distinguer clairement les prescriptions obligatoires des demandes dites « de confort ». Dans ce dernier cas, l'idée de prévoir une participation financière des fédérations est une piste intéressante, qui atténuera sûrement les prescriptions inutiles. Parallèlement, donner un rôle accru à la CERFRES est une démarche cohérente. Il apparaît nécessaire que les élus locaux puissent avoir un certain poids dans l'établissement des normes. La volonté, portée notamment par l'ANDES, d'adapter et d'ajuster les dispositions en fonction du territoire et de leur besoin me semble sage. D'ailleurs, je tiens à relayer les récentes critiques de cette association concernant les projets disproportionnés des ligues professionnelles de basket-ball et volley-ball pour renforcer la publicité dans les salles lors des matchs. Néanmoins, notre objectif doit être non pas d'entrer dans un rapport de force avec les fédérations, mais plutôt d'approfondir le dialogue pour définir les nouvelles dispositions à appliquer. Je tiens à saluer et à remercier mes collègues auteurs de cette proposition Le texte permettra, j'en suis certaine, une prise de conscience, notamment de la part des fédérations, car nous devons faire des collectivités des acteurs, et non plus de simples payeurs, de la création et de l'entretien des équipements sportifs. Je soutiendrai donc cette résolution. La parole

dans sa philosophie générale, la présente proposition de résolution est plus que bienvenue au regard des 400 000 normes qui s'imposent, entre autres, aux collectivités territoriales et qui régissent les 250 000 équipements sportifs qui maillent notre territoire. Dès 2013, Jean-Claude Boulard et Alain Lambert avaient été chargés d'une mission sur la lutte contre l'inflation normative par le gouvernement de l'époque. Leurs travaux ont souligné la préoccupation des collectivités face à la multiplication des normes auxquelles elles doivent se conformer. Le rapport de la mission commune d'information du Sénat sur le sport professionnel et les collectivités territoriales, présidée par Michel Savin, ainsi qu'un ainsi qu'un rapport de l'IGAS datant de 2015 arrivaient à un constat voisin. Les collectivités territoriales sont de très loin les premiers financeurs du sport ; je sais l'importance qu'accordent nos élus aux problématiques de sécurité et d'accessibilité. Mais, parallèlement, je n'ignore pas que ce corpus normatif n'est pas sans poser de problèmes et est généralement vécu comme une contrainte, du point de vue tant de la compétitivité que de la mise aux normes. Une consolidation apparaît donc nécessaire ; je pense que nous nous entendons parfaitement sur ce point. Conscient de l'impact de certaines règles édictées par les fédérations et à l'écoute de la préoccupation des élus territoriaux, le ministère des sports a déjà renforcé le rôle de la CERFRES, en affermissant celui des collectivités territoriales. Aujourd'hui, la CERFRES est ainsi composée d'un tiers de représentants des collectivités territoriales, d'un tiers de représentants de l'État et d'un tiers de représentants du mouvement sportif. Son président est par ailleurs élu au sein des membres du collège des collectivités territoriales. Aujourd'hui, dans le projet de résolution qu'il présente, le Sénat entend renforcer le rôle de la CERFRES, en préconisant simultanément des améliorations de son fonctionnement, mais aussi un renforcement de son champ de compétences. Ces propositions d'évolution sont pertinentes. Elles correspondent aux évolutions discutées et souhaitées au sein même de cette commission. Il est à noter que cette proposition de résolution s'inscrit pleinement dans la démarche du Gouvernement. Comme vous le savez, le Premier ministre a confié, au début de 2018, à MM. Lambert et Boulard une nouvelle mission relative à la simplification des normes les règles relatives aux équipements sportifs seront évaluées. Les propositions contenues dans cette résolution sénatoriale consolident donc la démarche générale de simplification, fondée sur une évaluation partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Je souscris à la philosophie des propositions d'ordre réglementaire. Je souhaite qu'elles inspirent la réforme que nous conduirons dans cette matière. Plus précisément, concernant le fonctionnement de la CERFRES, intégrer des élus d'intercommunalités et de communes rurales au sein du collège des élus permettra en effet d'en renforcer la représentativité et de mieux prendre en compte les différentes spécificités territoriales. à trois mois du délai d'examen des projets de règlement permettra de consolider les échanges entre les différents acteurs et facilitera la prise en compte de l'avis des élus quant à l'impact des règles proposées.

Cela tend à démontrer la réussite de la concertation entre les différents acteurs au sein de la CERFRES. Il est par ailleurs important de rappeler que, en sus de l'existence de cette procédure, un membre du CNEN participe aux travaux de la commission et que la CERFRES

la possibilité de réexaminer des règlements fédéraux après un délai de mise en oeuvre, afin d'en faire l'évaluation et de pouvoir tenir compte de l'expérience des collectivités territoriales, reprend l'une des réflexions menées lors de la réunion de cette La mise en oeuvre de cette procédure permettrait en effet, en prenant en compte l'expérience du terrain, de réévaluer l'impact d'un règlement et, potentiellement, d'en rediscuter la mise en oeuvre avec la fédération émettrice. Le pouvoir d'autosaisine de la commission est aussi une piste de réflexion souhaitée au sein de CERFRES. Celle-ci, qui regroupe les différents acteurs concernés, semble en effet le lieu de concertation privilégié pour discuter d'évolutions réglementaires pouvant avoir un impact positif sur le fonctionnement des équipements sportifs. Il est à noter que la CERFRES a déjà été à l'initiative de deux modifications réglementaires récentes ayant eu un impact significatif sur les finances locales la diminution du nombre de vidanges obligatoires dans les bassins de natation et la modification du décret « buts ». Permettre à la CERFRES de se saisir systématiquement des labels d'ordre commercial des ligues professionnelles et autres recommandations, les « normes grises ou de toute règle ayant un impact sur l'exploitation des équipements va aussi dans le sens d'une démarche générale de simplification fondée sur une évaluation partagée avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment de la prise en compte des propriétaires des équipements. Ce sujet n'a cependant pas été discuté à ce stade avec le mouvement sportif et nécessiterait une concertation préalable. La disposition relative à la règle « prescripteur-payeur », envisagée, mais sans être proposée dans le projet de résolution, s'applique déjà en en partie dans le cadre des conventions de mise à disposition des équipements entre les propriétaires et les utilisateurs. Pour éviter un un risque de blocage du développement et de la sécurisation des activités sportives, il semblerait au préalable important d'en circonscrire le champ d'application en l'envisageant notamment pour les « normes grises

Elle rejoint également les évolutions qui étaient souhaitées par les acteurs de la CERFRES pour le renforcement de son action, soucieux de ne pas altérer le développement de l'offre de pratique sportive tout en préservant les finances locales. En outre, les mesures de renforcement préconisées pourraient également associer le positionnement de la CERFRES, intégrée comme sous-commission du Conseil national du sport depuis 2013.

Mesdames, messieurs les sénateurs, les propositions formulées dans cette proposition de résolution vont dans le bon sens, celui du dialogue et de la coconstruction nécessaires entre fédérations et collectivités. Le Gouvernement est très sensible à cette méthode. C'est aussi dans cette optique que le Premier ministre a lancé un groupe de travail Lambert-Boulard sur la maîtrise des normes applicables aux collectivités territoriales. Je suis persuadée qu'il saura prendre en compte vos propositions dans ses travaux. La discussion

la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Je mets aux voix la proposition de résolution.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses

procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur du débat disposera d'un temps de parole de dix minutes, y compris la réplique,

des conclusions du Conseil d'orientation des infrastructures, le COI, sur un sujet caractérisé depuis trop longtemps, il faut oser le dire, par les annonces et la fuite en avant, et par une technique bien connue en politique et bien éprouvée, qui veut que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ! La mission confiée au COI consistait donc à évaluer les besoins en termes de mobilité, à étudier les projets de transport sur tout le territoire et à les prioriser selon une grille comportant six critères d'évaluation environnement, mobilité pour tous-solidarité, qualité de vie-efficience, sécurité et sûreté, aménagement du territoire, enfin création de valeur socio-économique. Il s'agissait aussi de trouver des pistes de financement associées, en fonction des différents scénarios. Car avec une dette publique établie à 2 500 milliards d'euros à la fin de l'année 2017, soit plus de 95 % de notre PIB, il est plus que temps de céder enfin au réalisme, d'en finir avec les promesses qui n'engendrent que frustrations et déceptions, et donc de tenir compte de la contrainte financière. C'est également ce que préconise le rapport Spinetta, qui ne fait que renforcer les conclusions du COI. Partageant cette approche faite de rigueur et de pragmatisme, j'ai accepté d'être membre du COI, composé de dix élus locaux, nationaux et européens de différentes sensibilités politiques, et de six personnalités qualifiées. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de retrouver deux collègues sénateurs, Hervé Maurey et Michel Dagbert, ainsi que notre ancien collègue Louis Nègre, spécialiste de ces sujets.

ce rapport est guidé par une logique forte, qui vise à transformer en actes les intentions affichées. Si l'expression des politiques générales est admise par tous, en tirer les conséquences concrètes, en rupture avec les habitudes antérieures, est forcément plus délicat. Il n'est pas question de délaisser le ferroviaire ni de se désengager des territoires ruraux, comme on a pu l'entendre dire depuis la parution du rapport. Il n'est pas question non plus de ne maintenir que les lignes qui seraient considérées comme rentables ou susceptibles de l'être. Il est question, simplement, de mieux prioriser les dépenses de l'État le transport ferroviaire doit répondre à des besoins effectifs. Si l'on estime que l'on ne peut plus se permettre de maintenir un trafic qui ne serait pas suffisamment utile, il est bien évident qu'il faut trouver des modes alternatifs de transport permettant aux habitants de circuler le plus facilement possible. Le travail du COI a donc consisté à analyser une série de projets et leur coût, face aux crédits disponibles- j'insiste bien sur ce dernier

Nous avons discuté, fait des choix et proposé au Gouvernement trois scénarios, construits à partir du périmètre actuel des transports de l'État, dans tous les modes, excepté l'aérien qui sera traité dans le cadre des Assises de l'aérien. Trois scénarios l'un à 48 milliards d'euros, l'autre à 60 milliards d'euros et enfin le dernier à 80 milliards d'euros. C'est-à-dire que le COI a fait le choix de repousser plus ou moins loin dans le temps les grands travaux en les découpant, dans certains cas, en phases successives.

à partir de recettes existantes ou de nouvelles recettes à trouver. Ce scénario permet d'avancer les premières phases des grands projets les plus utiles et de réduire la saturation des principaux noeuds ferroviaires. Les projets sont ensuite poursuivis de façon progressive. L'effort est encore accru avec le troisième scénario, qui prévoit 80 milliards en vingt ans pour l'AFITF, soit 3,5 milliards d'euros par an à court terme d'ici à 2022, puis 4,4 milliards d'euros par an durant les dix années suivantes, et ensuite 4 milliards d'euros

d'une part, pour les collectivités territoriales appelées à cofinancer, d'autre part, pour l'État supposé être en mesure de dégager des moyens accrus.

Oui, il est absolument fondamental de traiter prioritairement les noeuds ferroviaires afin de rendre les gares plus efficaces et fiables, de décongestionner les accès aux principales gares et de préparer la création de lignes nouvelles, sous peine de contribuer encore plus à leur saturation. C'est une urgence et une priorité absolue. Les usagers ne savent pas toujours qu'un train à l'arrêt n'est pas forcément en panne et qu'il peut tout simplement être obligé d'attendre son tour. S'agissant des TGV, cet engorgement, ces retards ne sont pas admissibles. Il n'est pas non plus admissible que les TGV soient trop souvent à l'approche des gares, alors qu'ils sont conçus pour rouler à une vitesse bien plus élevée. La résorption des noeuds ferroviaires permettra aux TGV circulant de conserver leur vitesse optimale. À quoi sert-il d'avoir construit des lignes spécifiques si les TGV sont obligés d'y rouler à la vitesse de TER à cause des noeuds ferroviaires ? Les noeuds ferroviaires franciliens qui perturbent l'accès aux grandes gares franciliennes doivent être prioritairement décongestionnés, et pas seulement à Paris. On parle trop souvent- à tort selon moi-de Paris, qui aurait été privilégié. Il faut également traiter le noeud ferroviaire lyonnais, qui présente le plus grand caractère d'urgence. Mais aussi traiter les noeuds ferroviaires du nord de Toulouse et du sud de Bordeaux, Marseille et Nice, sans oublier- le rapport le précise d'ailleurs -d'agir rapidement sur des noeuds de plus petite ampleur.

Cette ouverture impose la mise à niveau de notre patrimoine ferroviaire, qui a commencé à se déliter avec la priorité accordée à la création de nouvelles lignes de TGV. C'est pourquoi le COI a insisté, au-delà des noeuds ferroviaires, sur le maillage du territoire, en préconisant la régénération des lignes de trains du quotidien et la rénovation des lignes ferroviaires existantes. Pour conclure, est-ce la fin de l'histoire pour les projets qui ne sont pas retenus par le Conseil d'orientation des infrastructures ? Bien sûr que non ! Le COI a rejeté très peu de projets. Dans la plupart des cas, il a simplement considéré que tel ou tel projet était moins prioritaire et pouvait attendre. Ces projets pourront donc être réexaminés dans le cadre d'une clause de revoyure. Le COI a fait des propositions en vue d'une programmation qui a vocation à être inscrite dans la loi d'orientation sur les mobilités. Il appartient maintenant au Gouvernement de décider des suites qu'il entend donner à ces propositions, puis de les traduire dans un projet de loi soumis à la représentation nationale. Je vous remercie,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, lors de son discours du 1 juillet à Rennes, le Président de la République a souhaité que la politique des mobilités se recentre sur les préoccupations premières de nos concitoyens et de nos entreprises les transports du quotidien, la lutte contre la congestion des grandes agglomérations, l'accès à l'emploi et aux services dans les territoires, l'optimisation de nos systèmes logistiques. Il a voulu également que cette réforme s'engage dès le début du quinquennat. Les besoins de nos territoires, de nos concitoyens, de nos entreprises, évoluent, vous le savez, rapidement, et le secteur des transports doit contribuer activement à la transition écologique, dans un contexte marqué par les contraintes qui pèsent sur les capacités financières des pouvoirs publics : sur celles de l'État et, j'en suis consciente, sur celles des collectivités. L'État et les collectivités territoriales doivent donc anticiper et accompagner ces évolutions en révisant en profondeur leurs stratégies et leurs modes d'action. En effet, pour ne prendre que l'exemple du ferroviaire qui sera au coeur de nos échanges pendant les prochains jours, si l'inauguration de quatre lignes à grande vitesse au cours des deux dernières années peut être un légitime motif de satisfaction, voire de fierté, qui peut se satisfaire de la dégradation continue de nos infrastructures de transports, des 5 300 kilomètres de notre réseau ferré sur lesquels nos trains circulent au ralenti et ne sont plus à même de répondre aux besoins des usagers ? Il y a donc urgence à revisiter nos choix d'investissement et, là où des promesses non financées ont longtemps créé de faux espoirs, abîmé la confiance de nos concitoyens dans les engagements de l'État, nourri le sentiment d'abandon de nombreux territoires, nous voulons leur proposer un nouveau cadre d'action et de programmation tourné vers les besoins du quotidien, équilibré en ressources et en dépenses. Ce besoin de changement, votre Haute Assemblée l'appelle de ses voeux depuis plusieurs années. Ce besoin de changement, nos concitoyens l'ont exprimé avec impatience dans les ateliers territoriaux des Assises nationales de la mobilité. Cette impatience, celle dont vous êtes également les témoins dans vos territoires, je la comprends, je la partage et je mesure l'urgence de lui apporter une réponse, au risque de voir se creuser les fractures sociales et territoriales. Le Gouvernement s'est donc employé à ouvrir une page nouvelle, faite d'écoute, de cohérence et de sincérité. C'est le sens de la mise en place en septembre dernier du Conseil d'orientation des infrastructures, présidé par Philippe Duron. Ce conseil, je l'ai souhaité composé de femmes et d'hommes en prise directe avec les besoins des territoires et de nos concitoyens. J'ai souhaité qu'il représente la diversité des collectivités territoriales. J'ai souhaité que ses travaux puissent s'enrichir de la diversité des horizons tant professionnels que politiques de ses membres. Permettez-moi de saluer, devant vous, l'engagement de vos collègues qui ont activement contribué aux travaux du COI : Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, Gérard Cornu, que je remercie d'être à l'initiative de ce débat, et Michel Dagbert. La mission confiée était ardue, ils n'ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour réussir cette ambition collective. Au final, c'est bien à l'unanimité des membres du COI que le rapport qui m'a été remis le 1 février dernier a été adopté. Il débouchera, vous le savez, sur une loi de programmation qui vous sera présentée dans les prochaines semaines, et répondra ainsi à la première recommandation formulée par la commission des finances du Sénat en septembre 2016

sur la base des travaux d'une commission permanente composée d'élus nationaux, locaux et d'experts, qui sera ensuite chargée d'examiner tous les ans l'avancement des projets programmés et de proposer, le cas échéant, des ajustements

durant quatre mois d'un travail considérable qui fera date, ponctué par plus de cinq cents auditions. Ce rapport réinterroge de fond en comble notre politique d'investissements dans les infrastructures, en repartant d'une question simple et primordiale : à quels besoins devons-nous répondre en priorité ? ? Il propose trois scénarios. C'est là aussi le caractère inédit de ce travail : les membres du COI ont placé les besoins d'investissements face aux réalités des moyens que nous devons y consacrer. Le scénario Le scénario n° 1, à ressources constantes, permet juste de satisfaire les besoins d'entretien du patrimoine existant. Il fait donc preuve de sincérité en montrant ce qu'il est possible de faire à ressources constantes. Le scénario n° 2 permet de répondre aux priorités fixées par le Président de la République et nécessite d'affecter au secteur des transports des moyens supplémentaires significatifs, à hauteur de 600 millions d'euros par an.

Les trois scénarios, je le répète, ont le mérite de la cohérence. Ils mettent tout le monde face à la complexité et à la réalité de l'équation qui s'impose à nous. Quel que soit le scénario que nous choisirons, le rapport nous recommande un certain nombre de priorités. Je dois dire que j'y ai retrouvé beaucoup de mes convictions Elles répondent en effet toutes au coeur du combat que je mène pour les transports du quotidien. Il préconise tout d'abord l'entretien et la régénération des réseaux existants. Chacun a en tête les innombrables exemples d'un réseau, qu'il soit ferroviaire, routier ou fluvial, qui marque des signes de fatigue par manque d'entretien. Ce n'est tout simplement plus tenable. Il s'agit là d'un besoin que je qualifierai d'élémentaire, de vital ! L'autre priorité mise en avant, à laquelle je sais que vous êtes particulièrement attentifs, est le désenclavement de tous nos territoires. Voilà un exemple d'une politique d'infrastructures qui ne tourne plus rond : c'est ce que je me dis quand, dans mes déplacements, je suis confrontée à des habitants, à des élus, qui désespèrent de voir la modernisation de certains axes routiers repoussée de contrat de plan en contrat de plan, de décennie en décennie, alors que ces chantiers sont pourtant indispensables ! Il ne s'agit pas de grands travaux, mais de contournements de bourgs, d'aménagements de sécurité, de créneaux de dépassement, indispensables pour relier correctement tout notre territoire. Je l'ai indiqué, je suis convaincue que ce désenclavement routier peut être achevé en l'espace d'une décennie.

La place du ferroviaire reste naturellement essentielle dans le désenclavement des territoires au travers des « petites lignes », terme impropre pour qualifier des lignes souvent essentielles aux besoins de mobilité de nombreux territoires. La dernière priorité est celle des mobilités douces, dont le vélo, bien sûr. Je me suis réjouie que le COI ait fait de ce mode de transport propre, extrêmement pertinent sur de nombreux trajets du quotidien, un élément central d'une politique d'équipement. Cela participe d'une prise de conscience en faveur de laquelle je milite beaucoup. Quant aux projets d'infrastructures tant discutés, le COI a apporté au débat une vision nouvelle, qui me semble extrêmement novatrice et utile. En effet, sur bon nombre de projets, le débat ne peut se résumer à la question de faire ou de ne pas faire. Le rapport souligne parfaitement qu'un grand projet peut très bien se réaliser et répondre à nos priorités, selon le rythme et le phasage qu'on lui donne. Le rapport du COI ouvre, je le souhaite, une nouvelle page et une nouvelle approche dans nos choix d'investissement. Il nous donne les outils nécessaires pour sortir des impasses financières et politiques sans renoncer à notre ambition collective de répondre aux besoins de mobilité de nos concitoyens. En effet, il ne s'agit pas de dépenser moins, de faire des économies. Nous aurons même à investir plus, à engager davantage de moyens pour nos infrastructures ! Mais l'enjeu est aussi et d'abord d'investir mieux, c'est-à-dire de faire des choix pertinents pour nos concitoyens, de répondre à leurs besoins, de telle sorte que chaque euro investi soit le plus utile possible. Le Gouvernement fera bientôt connaître ses choix. Il vous appartiendra de débattre de ces investissements et d'une programmation sincère de nos infrastructures pour les prochaines années, à la fois pour améliorer le quotidien de chacun, mais aussi pour la crédibilité de la parole publique. Ce débat, nous l'engageons aujourd'hui, et je m'en réjouis, car je suis convaincue qu'il viendra très utilement compléter les nombreuses consultations que j'ai engagées depuis le mois de février et qui m'ont permis d'échanger directement avec certains d'entre vous. À l'aune de ce débat, consciente que de vos travées trouveront à s'exprimer les légitimes attentes des territoires que vous représentez, je veux vous rendre attentifs au défi que nous avons à relever ensemble, celui de définir une stratégie ambitieuse, réaliste et cohérente, car, pour reprendre les propos de vos collègues Hervé Maurey et Louis-Jean de Nicolaÿ dans leur rapport de mai dernier, « si chacun de ces projets, pris individuellement, peut paraître fondé, leur agrégation ne répond à aucun moment à une stratégie d'ensemble véritablement réfléchie et intégrée C'est cette stratégie que je souhaite pouvoir construire avec vous ! Je rappelle

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, 105 kilomètres, c'est la distance de la ligne LGV Bordeaux-Dax que le rapport Duron condamne. Ce projet, qui avait été étudié et débattu dans le cadre du Grand projet du Sud-Ouest, le GPSO, a été repoussé à un horizon incertain, alors qu'il avait été validé par le territoire. Il ne s'agit pas d'une discussion technocratique, car le GPSO bénéficie d'un important soutien populaire, comme l'atteste un récent sondage IFOP Sud-Ouest 80 % des sondés en Nouvelle-Aquitaine sont favorables à la ligne Bordeaux-Toulouse et 78 % à la ligne Bordeaux-Dax. Cette ligne Bordeaux-Dax est le maillon essentiel de l'axe ferroviaire du sud-ouest de l'Europe ; c'est « le » premier maillon de la future connexion du réseau ferré français au réseau espagnol. Qu'on ne s'y trompe pas, l'axe ferroviaire Paris-Bordeaux-Valladolid-Madrid est considéré comme l'un des axes stratégiques du réseau européen pour relier la péninsule ibérique au reste de l'Europe par la façade atlantique, tant pour le fret que pour le trafic voyageurs. Les temps de parcours compétitifs, l'augmentation du nombre de dessertes ferroviaires constituent de réels gains de performances. À l'échelle de la France, GPSO place Pau sous la barre des 4 heures pour rallier Paris, seuil essentiel pour le report modal de plus de la moitié des passagers de l'avion vers le rail. D'autant plus que la ligne Dax-Espagne est envisagée comme une solution de transport écologique et durable en réponse au trafic de lourds et aux 44 millions de tonnes de marchandises qui franchissent chaque année la frontière entre la France et l'Espagne. Seule la ligne complémentaire à l'offre TER au sud de Bordeaux rendra possible l'augmentation de capacité nécessaire au développement du fret ferroviaire de Bordeaux à Hendaye. Veuillez conclure ! Madame la ministre, quelles perspectives envisagez-vous dans la future loi d'orientation sur les mobilités pour la ligne LGV Bordeaux-Dax ? J'invite les

S'agissant plus précisément du trajet Bordeaux-Dax, le COI a proposé de différer le financement de la ligne à une étape ultérieure, mais également de sécuriser le tracé prévu, qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. publique. Sans attendre la réalisation de ce projet, il convient aussi d'étudier avec SNCF Réseau les améliorations concrètes pouvant être apportées aux lignes existantes, les reports modaux, notamment pour les poids lourds, ne devant pas attendre la mise en service de la future ligne à grande vitesse. Comme vous le savez, les collectivités territoriales ont également proposé de travailler sur des sources de financement complémentaires.

Pour autant, nos concitoyens sont habitués à ce qu'on leur donne à fois la température qu'il fera demain et la température ressentie ! Une fois de plus, le constat est amer pour les élus des territoires à la suite de la publication du rapport, puisque nous pourrions superposer plusieurs cartes : celle des déserts médicaux, celle des fermetures de classes dans les secteurs ruraux, celle des fermetures de services publics et, enfin, celle des lignes dites « non rentables » qui pourraient être appelées à disparaître ! Mon intervention vise une fois de plus à vous alerter sur l'indispensable desserte des villes moyennes par le rail. Nos collègues élus en charge des collectivités autorités organisatrices de transport s'attachent à maintenir un maillage territorial digne de ce nom : ce serait un très mauvais signal que de venir fragiliser leurs efforts visant à assurer la mobilité pour tous. Cela peut se traduire de différentes manières. J'en veux pour exemple le renoncement à l'électrification de la ligne Rang-du-Fliers-Amiens ou encore la menace d'une moindre desserte TGV TGV des villes de Lens et de Béthune dans mon département. Madame la ministre, comment faire pour que nos villes moyennes bénéficient, demain encore, d'une connexion au réseau grande vitesse qui fait la fierté de la France ? La parole est à Mme la ministre.

: les politiques en matière d'infrastructures menées au cours des dernières années, en privilégiant les lignes à grande vitesse et la réalisation de nouvelles lignes à grande vitesse, accentuent la métropolisation de notre pays. Elles ont laissé de côté

accorde la priorité à l'entretien et à la modernisation des réseaux existants, au maillage et au désenclavement routier du territoire, au maintien d'un réseau dit « classique » de qualité et, bien sûr, à la poursuite du développement des lignes à grande vitesse, mais selon un calendrier cohérent et compatible avec les ressources que l'on pourra ou que l'on voudra y consacrer. Dans ce cadre du développement des lignes à grande vitesse, il n'est en aucun cas question de modifier le modèle du TGV. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, depuis le lancement de l'aventure qu'est le le modèle qui a été retenu dans notre pays est celui d'un TGV non seulement qui dessert les métropoles reliées par les lignes à grande vitesse, mais aussi qui poursuit son parcours pour assurer la desserte des villes moyennes.

des gouvernements successifs pour imposer le tout-TGV et négliger totalement, depuis des années, les TER et Intercités ? Ces dernières années, en effet, la SNCF a investi en crédits d'études beaucoup de temps et d'argent sur des projets de LGV, je pense à la ligne Limoges-Poitiers -et ne se réaliseront malheureusement jamais, au détriment des trains en activité. Je peux en témoigner à titre personnel comme d'autres qui, deux fois par semaine, utilisent la ligne Intercités POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, laquelle impacte directement

son aspect relatif à l'aménagement du territoire, qui demeure essentiel à mes yeux. Dans cette perspective, il faut sûrement optimiser le fonctionnement des LGV. Mais faut-il ouvrir de nouvelles lignes- à l'exception peut-être, dans un premier temps, de quelques-unes, comme celle de Nantes doit être aménagée en contrepartie de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, voire celle de Toulouse -ou privilégier la rénovation des TER et Intercités, indispensables au maintien de la vie et de l'activité de nos territoires ? Élu de l'ancienne région Limousin, je préconise la seconde solution, plus empirique, plus pragmatique à mettre en oeuvre. Pour assurer la continuité entre Paris et les territoires, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre notion de service public et rentabilité, mais en tenant compte des nécessités de l'aménagement du territoire, et en procédant à une large concertation, non pas seulement entre l'État et la SNCF, mais aussi avec les collectivités territoriales. C'est pourquoi, madame la ministre, je souhaite, au-delà de ce débat, que la réforme de la SNCF annoncée par le Gouvernement réussisse et permette de maintenir les TER et les Intercités. Ne laissons pas mourir ce patrimoine qui constitue le maillon fort du désenclavement, de l'aménagement du territoire, et revitalisons-le dans l'intérêt de la Nation.

La réforme ferroviaire est partie intégrante de la stratégie de mobilité pour notre pays, au même titre que la loi d'orientation des mobilités, avec une priorité : la qualité du service rendu aux usagers et aux territoires. Oui, il faut le dire, nous avons délaissé des pans entiers de notre réseau ferroviaire classique, parfois dans l'espoir de voir arriver une ligne à grande vitesse, nécessairement à long terme. terme. Je vous le confirme, nous souhaitons inverser cette tendance. Par exemple, la ligne POLT, qui vous est chère, bénéficiera dans les décennies à venir de très lourds investissements pour régénérer l'infrastructure, renouveler le matériel roulant,

puissent renouer avec la noblesse qui était la leur à une époque où le Capitole était le train le plus rapide de France. Il faut absolument sortir d'un schéma dans lequel

réforme ferroviaire, ma priorité est bien que notre système ferroviaire réponde d'abord aux besoins de transports du quotidien de nos concitoyens.

Je rappelle qu'en septembre 2016, l'État, la SNCF, la région Île-de-France, la région Grand Est, le département de l'Aube et les villes de ce département qui sont traversées par une ligne ferroviaire ont signé un protocole et commencé à financer les travaux.

quelle est la nature de l'engagement du Président de la République en faveur d'un aménagement du territoire équilibré ? La ville de Troyes est la seule agglomération qui n'est pas raccordée par un train électrifié ! Pour tenir

la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a déjà pu entendre M. Duron sur les scénarios du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. En termes d'aménagement, de maillage et de desserte du territoire, je voudrais juste partir d'un cas particulier pour mieux montrer l'attente de certains départements en matière d'équité territoriale et de désenclavement. Certaines agglomérations bénéficient d'un statut de métropole de premier plan avec un TGV qui dessert la capitale. Pour d'autres, la réalité des temps de trajet ne cesse de se dégrader. Si je prends l'exemple de la zone du grand Massif central, et plus particulièrement de Clermont-Ferrand, le parcours en train aujourd'hui 30 et 4 heures quand tout va bien. Mais les différents aléas que vivent les usagers montrent que ça ne va pas toujours bien ... Sur une carte isochrone, Clermont se retrouve au sud de Marseille, ce qui en fait la métropole la plus éloignée de la capitale Sur la ligne Paris-Clermont, les derniers travaux d'entretien importants datent de 1990, avec l'électrification de la ligne. On en mesure aujourd'hui les carences et les conséquences, que ce soit en matière de temps de parcours, de régularité ou de confort à l'intérieur du train. Ce mode de transport souffre d'une absence de communication quant aux programmes et calendriers de travaux en cours et à venir sur ces lignes d'équilibre du territoire. On nous parle depuis longtemps déjà d'un changement possible de matériel ou de temps de parcours améliorés, mais nous avons toujours l'impression de décisions repoussées. ailleurs, la mobilisation pour un TGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon, dit POCL, destiné avant tout à anticiper l'éventuelle saturation de la ligne Paris-Lyon, a pendant un certain temps capté l'attention et les efforts, et a mis de côté les nécessaires entretiens ou améliorations des lignes structurantes. Ma question est donc double.

qui contribue fortement à l'intérêt socio-économique de cette nouvelle ligne, interviendra beaucoup plus tard que ce qui était envisagé grâce aux

que, sans attendre- or c'est bien l'exemple d'une ligne où l'on a trop attendu les TGV -, des améliorations substantielles puissent être apportées sur la ligne classique.

ces travaux d'amélioration rapide de la ligne existante seront bien pris en compte et programmés en donnant de la lisibilité et de la visibilité à l'ensemble des élus et des citoyens intéressés par sa modernisation.

Ce que demandent les Finistériens, c'est de disposer de conditions de transport qui les rapprochent des principaux centres de décision nationaux et européens, et qui permettent à la pointe bretonne de se développer. Contrairement à ce que semblent penser les membres du Conseil d'orientation des infrastructures, la Bretagne ne se résume pas à un axe Rennes-Nantes. Alors, après avoir rapproché Rennes de Paris grâce à la nouvelle ligne à grande vitesse, il faut maintenant rapprocher Brest et Quimper de Rennes. Pour apaiser la légitime colère des Finistériens après la publication de ce rapport qui les oublie, et à la suite de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dames-des-Landes, le Gouvernement a confié une mission- encore une ! -à M. Rol-Tanguy, cette fois sur les mobilités du Grand Ouest. Je forme le voeu, madame la ministre, que cette mission ne soit pas une nouvelle manoeuvre dilatoire, mais qu'elle permette au contraire au Gouvernement de concrétiser enfin cet objectif crucial des 3 heures en train entre Brest et Quimper, d'une part, et Paris, d'autre part, objectif encore rappelé par les collectivités territoriales bretonnes dans le pacte d'accessibilité de la Bretagne qu'elles proposent à l'État.

soutenir les collectivités locales dans la préparation d'une stratégie de desserte du Grand Ouest, en tenant notamment compte des enjeux de desserte au sein de la Bretagne. Cette stratégie qui sera présentée avant l'été,

l'incompréhension des élus locaux, notamment dans mon département, l'Isère, au sein de la métropole grenobloise. Cette incompréhension, je ne suis pas loin de la partager, surtout après les engagements pris lors des Assises nationales de la mobilité, de prioriser les mobilités du quotidien et, notamment, de doter les aires métropolitaines « d'un réseau ferroviaire capable d'apporter une réponse à la saturation et à la congestion routière Or ce rapport témoigne, je dois le dire, d'une absence totale de prise en considération des enjeux s'attachant, en particulier, à la desserte ferroviaire de l'aire métropolitaine grenobloise. Les enjeux de cette aire sont pourtant multiples. répondre aux objectifs d'attractivité et de rayonnement d'un territoire qui est le deuxième pôle de recherche scientifique à l'échelle nationale. Par ailleurs, ce sont 750 000 habitants et 320 000 emplois qui souffrent d'une réelle insuffisance de l'offre ferroviaire et d'une qualité de service dégradée, caractérisée notamment par un manque de fiabilité qui pèse sur le quotidien des usagers, tout particulièrement sur la ligne Grenoble-Lyon, première liaison ferroviaire de la région en termes de nombre de voyageurs et qualifiée de « malade » dès 2011 par Guillaume Pepy.

de la ligne Grenoble-Paris, cette liaison ayant vocation à s'inscrire dans le cadre des « grands projets de liaisons entre métropoles », un des objectifs stratégiques identifiés par le rapport deuxièmement, l'identification de l'étoile ferroviaire grenobloise comme territoire prioritaire et volontaire de développement d'un « RER » métropolitain. Aussi, madame la ministre, nous souhaiterions être éclairés sur la manière dont le Gouvernement entend répondre à ces enjeux dont j'espère avoir suffisamment souligné l'importance capitale pour la métropole grenobloise, le département de l'Isère et, au-delà, la région Auvergne-Rhône-Alpes. La parole est à Mme la ministre. S'il est

des noeuds ferroviaires lyonnais et grenoblois, par le nombre et la diversité des circulations- TER, TGV, trains de fret -, et par les caractéristiques techniques de la ligne, avec un temps de parcours qui ne peut clairement pas être considéré comme satisfaisant. Une première enveloppe de 20 millions d'euros est prévue dans le contrat de plan 2015-2020 entre l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour réaménager le plan de voies à Saint-André-le-Gaz, qui constitue un point névralgique du réseau. Cela permettra d'améliorer, à la fois, les liaisons Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry.

de financement des infrastructures, et dresse toute une série de constats et de propositions. Parmi les constats figure celui du sous-investissement des pouvoirs publics qui, depuis trop longtemps, a conduit à l'obsolescence d'une partie du réseau et à des ralentissements portant atteinte à la performance même du service public. La concurrence voulue par les ordonnances n'est, à ce titre, aucunement une réponse, puisque la qualité du service proposé dépend principalement, aujourd'hui, de l'état des infrastructures. Si le rapport reconnaît que les sources de financement se sont raréfiées, il ne promet comme solutions nouvelles que celle qui consiste à faire payer davantage les usagers, ainsi qu'une reventilation de l'affectation des taxes, notamment la taxe La troisième priorité d'action définie par ce rapport est l'aménagement du territoire et la lutte contre les inégalités. À ce propos, la LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon est un véritable enjeu pour l'ouverture des territoires du Centre, du Massif central, du Roannais. de rapprocher Saint-Étienne de Paris avec une régularité améliorée et un allégement du trafic sur la ligne, actuellement saturée, reliant Lyon et Paris. Vous le savez, plus ce projet sera repoussé, plus les travaux le seront aussi. Ce n'est pas acceptable, car les femmes, les hommes et les entreprises n'ont pas besoin d'une chimère, mais d'une véritable ligne structurante pour leur territoire. Ce rapport se borne à proposer des trajectoires financières peu ambitieuses dans un contexte budgétaire particulièrement

affirme une priorité à l'entretien et à la modernisation de nos réseaux, c'est-à-dire aux transports de la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous devrions tous pouvoir nous retrouver autour de cette priorité.

et affirmer à cette occasion mon attachement à l'offre de liaisons cadencées à grande vitesse dans les Hauts-de-France, l'un des piliers de l'aménagement de notre territoire. La desserte TGV TGV constitue une véritable colonne vertébrale en termes de dynamique et de maillage territoriaux, qu'il convient de conforter tant pour la métropole lilloise que pour les autres grandes agglomérations de la région

C'est un projet essentiel pour la mobilité, l'attractivité et le développement économique du territoire. Alors qu'un certain nombre de projets sont reportés, le rapport Duron confirme l'intérêt de cette liaison et différents scénarios de réalisation y sont proposés. Madame la ministre, quel scénario allez-vous privilégier, et selon quel calendrier ? Ma deuxième question porte sur la desserte en TGV des gares dites « autres gares desservies par le TGV » dans les Hauts-de-France ... Je pense à Arras, Béthune, Dunkerque, Douai, mais aussi à Valenciennes, dont vient de parler Aujourd'hui, force est de constater que le service et le cadencement sont dégradés. Faute d'investissements, notamment sur la mise en sécurité- je pense, par exemple, à la suppression des passages à niveau -, nous sommes passés à un temps de trajet d'environ 1 heure 30 pour relier Paris à Valenciennes il y a une dizaine d'années, à près de 2 heures aujourd'hui. Le risque est évidemment de décourager les voyageurs et, faute de voyageurs, de justifier la fermeture de ces lignes. Madame la ministre, quelle est la stratégie du Gouvernement pour cette desserte des capitales infrarégionales des Hauts-de-France ? Pouvez-vous nous confirmer le maintien de ces lignes TGV pour les villes moyennes ? Enfin, vous l'avez compris, il conviendra d'engager rapidement des travaux qui devront permettre de retrouver un cadencement acceptable. La

L'enquête, qui devait être lancée, mais avait été suspendue dans l'attente des réflexions sur la programmation des infrastructures, pourra être conduite,

Je pourrais vous dire qu'il est toujours un peu contrariant de devoir investir pour retrouver les temps de parcours qu'on connaissait précédemment. Qu'il puisse y avoir des défauts d'entretien et de modernisation, je peux le comprendre, mais qu'il faille dépenser plus pour avoir le même temps de parcours peut nous conduire à nous interroger. Néanmoins, je vais demander à SNCF Réseau de me donner des explications, dans l'objectif de retrouver une desserte performante de ce territoire.

grande vitesse Grand Est en 2007, après de longs débats, la gare de Lorraine a été finalement implantée au milieu des champs, à Louvigny. Elle est surnommée par les Lorrains la gare « colza » ou « betteraves »- selon les goûts ! -en raison de son emplacement, certes équidistant de Metz et de Nancy, mais surtout déconnecté de toute liaison avec le réseau régional, notamment la ligne TER nord-sud entre Nancy et Metz, qui est structurante pour le sillon lorrain tout entier jusqu'à Luxembourg. La semaine dernière encore, j'étais en réunion à Nancy avec un intervenant de Poitiers,

Nancy. Ces situations sont également fréquentes dans d'autres lieux où les gares ne sont pas connectées au réseau TER. Maintenir cette gare à Louvigny relèverait d'une conception passéiste des lignes à grande vitesse, à l'heure où les transports doivent être envisagés, comme le et vous-même le proposez d'ailleurs, dans une logique de complémentarité et d'intermodalité des liaisons. Ainsi, l'ancienne région Lorraine est la seule des trois composantes de la nouvelle région Grand Est à ne pas avoir de gare TGV interconnectée à son réseau régional. Christian Eckert, alors secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics, a permis qu'une part non négligeable de ressources issues de la TICPE, estimée à 20 millions d'euros par an, soit fléchée à l'échelle régionale pour financer ce projet, profitant d'un dispositif européen qui le permet. Pourtant, la majorité régionale, très discrète sur le sujet, semble vouloir privilégier d'autres projets ferroviaires sans rapport avec une LGV. Madame la ministre, je souhaiterais connaître vos intentions sur ce sujet et savoir si la modification de l'implantation de la gare pourrait être confirmée dans la loi de programmation, afin que les financements envisageables soient enfin affectés à ce projet nécessaire aux mobilités du XXI siècle dans le Grand Est. La parole est à Mme la ministre. Vous le savez, monsieur le sénateur, l'ensemble du foncier nécessaire à la réalisation de la gare et de ses accès a été acquis, et des mesures conservatoires ont été prises lors de la réalisation de la première phase de la LGV est-européenne.

Il a été décidé que le conseil régional de Lorraine, en lien avec SNCF Réseau, assurerait la maîtrise d'ouvrage de la gare TER-TGV de Vandières. La part attendue de l'État s'élève à 30 millions d'euros dans le cadre de la convention de la deuxième phase de la LGV Est. Mais, à ce jour, aucun crédit n'a été budgété en ce sens. Le projet a fait l'objet- je veux le rappeler -d'un référendum régional organisé en février 2015 par le conseil régional de Lorraine, qui a conduit à un rejet. Je Je tiens à vous redire que le foncier est là et qu'il est disponible, mais qu'il revient aux collectivités de décider de l'intérêt ou non de réaliser cette gare, en tenant compte

Ce territoire, qui compte 17 millions d'habitants, soit 25 % de la population française, ne cesse d'attendre ... que ses besoins en mobilité soient pris en compte.

Nous vous avons rappelé l'importance de cette ligne pour la desserte et le désenclavement de notre territoire. Je tiens de nouveau à rappeler, comme cela vous a déjà été dit, que Clermont-Ferrand est la capitale régionale la plus éloignée de Paris en temps de transport ferroviaire.

la ministre, vous avez été rassurante. Vous nous avez certes rappelé que la rentabilité socio-économique du projet POCL était étroitement liée au doublement de la ligne Paris-Lyon.

que vous étiez favorable à la tierce expertise et que vos services allaient contacter les trois régions concernées afin de faire le point sur le plan de financement. Je vous confirme ici, dans cet hémicycle, que les trois présidents de région tiennent fortement que vous étiez pour la poursuite des travaux de l'observatoire de la saturation ferroviaire de la ligne Paris-Lyon et que, dès à présent, la ligne SNCF actuelle serait améliorée et rénovée afin que, de Paris, l'on puisse rejoindre Clermont-Ferrand en moins de 3 heures. Pourriez-vous, madame la ministre, nous confirmer ces points essentiels ?

projet. J'ai également dit qu'il ne fallait pas obérer l'avenir et se priver de la capacité de réaliser ultérieurement ce projet. Mais j'ai insisté, et je veux le répéter ici, sur le fait que ces réflexions ne doivent pas nous faire oublier la nécessité d'améliorer rapidement la ligne existante entre Paris et Clermont-Ferrand, ce qui sera le cas avec la livraison du nouveau matériel qui équipera cette ligne. Je le disais, les offres nous ont été remises le 15 mars dernier, avec l'objectif d'une couverture numérique de cette ligne dans les meilleurs délais, donc d'ici à la fin de 2018, au travers d'un schéma directeur en cours de discussion qui permettra de recenser les aménagements d'infrastructures utiles pour améliorer la performance du service ferroviaire sur cet axe. J'attends ce schéma directeur

qui souhaitait vous interroger sur la réalisation de la desserte ferroviaire de l'EuroAirport Bâle-Mulhouse. Ce raccordement vise à assurer un accès direct à l'aéroport par les trains régionaux avec, aux heures de pointe, six trains par heure en provenance et à destination de Bâle, et quatre trains par heure en provenance et à destination de Mulhouse. En plus de renforcer l'attractivité de l'EuroAirport, ce raccordement offrira une alternative à la route et contribuera à désengorger l'A35, qui connaît une forte fréquentation aux heures de pointe. Alors que ce projet a connu des avancées récentes avec la signature d'une déclaration d'intention commune entre la région Grand Est et les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de Soleure, laissant présager un début de travaux à l'horizon 2020, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures semble remettre en cause ce projet dans au moins deux des trois scénarios envisagés. En effet, dans deux d'entre eux, l'État ne participerait pas au financement de l'infrastructure, ce qui compromettrait l'équilibre financier du projet et sa réalisation à terme. Si nous comprenons la nécessité budgétaire qui conduit l'État à faire des choix répondant aux urgences du quotidien, il ne faut pas négliger ce projet qui présente à la fois un intérêt environnemental, en permettant de proposer une alternative à la route, et une dynamique transnationale de développement économique. côté suisse, la phase de consultation pour l'étape d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 2030-2035, en cours, a bien pris en considération le raccordement ferroviaire. Alors qu'il appartiendra au Parlement fédéral de confirmer cet engagement, il est capital pour la poursuite du projet que l'État français donne des garanties sur ses engagements et envoie, dès aujourd'hui, un signal fort à la Confédération helvétique en confirmant sa volonté de terminer les études et l'enquête publique d'ici à 2021 et de réaliser le projet sur la période 2022-2027. Madame la ministre, quel avenir, quel calendrier et quel financement par l'État envisagez-vous pour la desserte ferroviaire de l'EuroAirport ? La parole est à Mme la ministre. Effectivement,

que le COI n'a pas jugé prioritaire à court terme. Je sais l'attachement des élus à ce projet transfrontalier, de même que celui des autorités suisses.

Je suis tout à fait prête à recevoir une délégation pour échanger sur l'intérêt de ce projet. Nous attendons, à l'heure actuelle, une étude socio-économique pour apprécier les gains de chacun des acteurs, à la fois en France, en Suisse et en Allemagne, liés à la réalisation de ce projet, ce qui pourrait préfigurer des clés de financement pour la réalisation ultérieure du projet. Continuons à discuter avec les autorités suisses et les élus concernés pour voir dans quelle mesure, dans le cadre des contraintes financières qui sont les nôtres, nous pouvons envisager la réalisation de cette infrastructure dont je suis consciente qu'elle est attendue localement. La parole

les liaisons entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne : « la démonstration n'a pas été faite de l'urgence d'engager ces aménagements dont les caractéristiques socio-économiques apparaissent à ce stade clairement défavorables » et « ces travaux [ ...] seront à engager après 2038 ».

Ainsi, on constatait en 2017 moins de la moitié du volume prévu en 2006. De même, les circulations de fret ferroviaire franco-italiennes ont été divisées par six depuis trente ans, malgré 1 milliard d'euros d'investissements entre Lyon-Dijon et Turin. Les analyses démontrent d'ailleurs que le réseau ferré existant offre la possibilité, moyennant quelques investissements, d'accroître considérablement cette offre de fret. Le rail pourrait ainsi accueillir les marchandises d'un million de poids lourds par an dans les Alpes. Pourtant, après la pause décrétée au début de l'été, le Gouvernement, soufflant le chaud et le froid, a prorogé la déclaration d'utilité publique de cinq années. Nous peinons donc à comprendre s'il souhaite ou non engager la réalisation de ce tunnel, dont chaque kilomètre coûtera 150 millions d'euros. Cela est d'autant moins compréhensible que, sans les accès français et italiens, il est impossible de rentabiliser un tel ouvrage dont le modèle économique est déjà plus qu'incertain. J'aurais tendance à dire que l'on met la charrue avant les boeufs. Enfin, alors que l'incertitude politique italienne pèse également sur le tunnel, ce double discours paraît d'autant plus curieux. Si la finalité est l'abandon du projet, autant éviter d'enfouir 10 milliards d'euros dans 57 kilomètres de galeries sous les Alpes Madame la ministre, pourriez-vous nous préciser la logique sur laquelle s'appuierait le maintien d'un tel projet ? La parole est à Mme la ministre.

S'agissant du tunnel, je voudrais rappeler qu'il a fait l'objet d'un traité, qui a été ratifié par le Parlement en France comme en Italie. Les travaux de reconnaissance de la section internationale sont désormais réalisés à plus de 75 %, avec plus de 23 kilomètres percés à ce jour. ce jour. Les travaux définitifs du tunnel devraient être lancés au cours de l'année 2018. Je rappelle aussi que, en raison de son caractère binational, le projet dispose d'un plan de financement tout à fait spécifique, puisqu'il est financé à 40 % par l'Union européenne et à 35 % par l'Italie. La France porte ce projet à hauteur de 25 %, ce qui n'est pas rien pour un projet de 2,5 milliards J'ai eu l'occasion de le dire, l'enjeu est bien que la réalisation du projet ne vienne pas peser sur les ressources de l'AFITF, au détriment des des projets d'une dimension plus « habituelle » ou, en tout cas, des projets qui sont utiles pour le quotidien de nos concitoyens. C'est dans cet état d'esprit qu'une réflexion a été engagée avec nos collègues italiens pour mettre en place une société de projet, qui tirerait ses ressources notamment des tarifications applicables sur les autoroutes et ne viendrait pas obérer les capacités de financement

Il est préférable d'attendre de constater la réalité de la remontée du trafic avant d'engager des travaux coûteux pour l'aménagement des accès. Le tunnel de base fait bien l'objet d'un traité international au

sur l'ampleur des investissements envisageables en matière de transports. Il réalisait alors une revue des projets, en oubliant néanmoins d'étudier certains projets d'envergure, je pense en particulier au Grand Paris Express. Mais toujours est-il que ce rapport accordait une place de choix aux projets de lignes à grande vitesse, les LGV. Selon lui, trois scénarios seraient envisageables. Le premier prévoit de ne pas affecter de ressources supplémentaires significatives à ces projets, et donc de maintenir la pause annoncée par le Président de la République en la matière. Les deux autres préconisent, à différents degrés, un accroissement des dépenses pour accélérer leur réalisation. Le 15 février dernier était présenté le rapport Spinetta adoptant des conclusions quelque peu différentes. Il préconisait, entre autres, la fermeture des petites lignes et l'arrêt du développement du réseau TGV. Il avançait alors que le réseau TGV pouvait être aujourd'hui considéré comme abouti et que la construction de toute nouvelle ligne serait donc contre-productive. Par ailleurs, la Cour des comptes soulignait déjà en 2014 que le modèle français du ferroviaire à grande vitesse était devenu non soutenable. Madame la ministre, au regard de ces deux rapports et de la position de la Cour des comptes, opterez-vous pour le choix du développement continu des grands projets de LGV ou confirmerez-vous la pause annoncée par le Président de la République ? Qu'en est-il notamment de certains grands projets, tels que l'interconnexion des LGV entre Massy et Valenton, indispensable au bon fonctionnement de l'interconnexion des TGV autour de Paris et aussi à celui du RER C ? Cette interconnexion, alliée la réalisation de la ligne 18 du Grand Paris Express, permettra une plus grande efficience de la gare TGV de Massy, ainsi qu'un lien facile entre celle-ci et l'aéroport d'Orly. La parole est à Mme la ministre.

avec une triple interrogation : quelle place pour le ferroviaire dans notre politique de mobilité, comment remettre sur pied le modèle économique du ferroviaire, comment préparer une ouverture réussie à la concurrence ? Les deux rapports traitent de sujets disjoints. Les réflexions de Jean-Cyril Spinetta sur les petites lignes ferroviaires n'ont pas vocation à être reprises, le Gouvernement ayant largement fait savoir qu'il ne suivrait pas ces recommandations. Les réflexions sur les projets de lignes à grande vitesse sont étudiées à la fois du point de vue de leur phasage et de leurs modalités de financement, sur la base des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Dans ce cadre, je voudrais tout de même souligner que les scénarios ne se distinguent pas seulement par les rythmes de réalisation des lignes à grande vitesse, mais aussi par leur capacité à répondre aux priorités qui ont été affirmées l'entretien et la modernisation des réseaux, la désaturation des noeuds ferroviaires et le maillage du territoire, au travers notamment de la réalisation et de la mise à niveau de nos infrastructures routières. routières. Selon les cas, des lignes à grande vitesse, dont certaines sont fortement attendues dans les territoires, peuvent être réalisées de façon phasée. Je peux vous confirmer l'importance, du reste pointée par le rapport, d'améliorer l'interconnexion des TGV. C'est ce qu'attendent notamment les élus du Grand ouest. C'est ce qui pourrait également être attendu autour de la gare de Massy. Ce dossier, qui a un « certain âge », pose des problèmes d'insertion, notamment environnementale, mais sur lequel il est utile de reprendre les travaux pour trouver une solution. Il pose un enjeu de connexion de tous nos territoires sans passer par Paris.

Mme Angèle Préville. Madame la ministre, la ligne à grande vitesse devant relier Toulouse à Bordeaux a été jugée prioritaire, et je m'en réjouis. Nous sommes pourtant loin de la mise en service prévue par le projet initial GPSO. Selon les envisagés, la durée des travaux pourrait varier entre dix et vingt ans. Même dans le scénario n° 1, le plus contraint, seule la section Agen-Toulouse serait réalisée. Si une chose est pourtant évidente, c'est bien que la région Occitanie ne peut pas attendre vingt ans. L'enjeu de la mise en service de la ligne Toulouse-Bordeaux est bien celui de sa temporalité. L'aire urbaine de Toulouse comporte 1,2 million d'habitants et accueille le siège mondial d'Airbus. Elle est la quatrième plus grande aire urbaine du territoire, avec une croissance de 1,5 % par an. À ce titre, je rappellerai une récente enquête de l'URSSAF qui montre que notre région a créé 28 000 emplois sur les cinq dernières années, soit quatre fois plus que la moyenne nationale. Cette attractivité indéniable se heurte pourtant à certains freins : un corridor routier saturé, des petites lignes menacées dans toute la région et le manque effectif d'une ligne à grande vitesse. Au travers de ce projet de ligne à grande vitesse, il est question d'équité territoriale d'un aménagement du territoire équilibré, afin qu'une région dynamique et vivante puisse continuer à se développer sans des freins qui finiraient par lui être préjudiciables. Malgré la LGV Paris-Bordeaux, le temps de trajet actuel entre Paris et Toulouse dépasse largement 4 heures, 4 heures 20. Comment admettre que Toulouse soit la seule grande capitale régionale qui ne soit pas reliée à Paris par une ligne à grande vitesse ? Il est clair que, face à de tels enjeux économiques et démographiques, le rail est une des clés du désenclavement de nos territoires. Les perspectives du scénario n° 3 interrogent sur les dépenses à prévoir dans un cadre financier et budgétaire restreint. Pour atteindre ce scénario, qui est- vous vous en doutez -celui que nous appelons de nos voeux, et pour mieux répondre aux attentes des territoires, quels financements peut-on imaginer ? La Merci de votre réponse, madame la ministre. le projet GPSO, mais on pourrait aussi parler de la ligne Montpellier-Béziers-Perpignan et de l'autoroute Toulouse-Castres.

à la fois des lignes à grande vitesse qui sont attendues, en l'occurrence deux pour la région Occitanie, et des besoins de désenclavement des territoires. Je pense au cas de Castres, où le maintien d'entreprises importantes sur ce territoire est conditionné à l'amélioration de la desserte routière à la remise à niveau des infrastructures nécessaires pour les trains du quotidien. C'est bien l'ensemble de ces besoins qu'il nous faut prendre en compte, et c'est tout le sens de la démarche du Conseil d'orientation des infrastructures. Vous l'avez rappelé, selon les scénarios,

oublié de moderniser ou, en tout cas, qui n'avait pas été modernisée dans les temps. Le calendrier qui sera finalement retenu fait l'objet de travaux avec les collectivités concernées des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, qui ont réfléchi à de nouvelles sources de financement, à l'instar de ce qui peut exister en Île-de-France avec la Société du Grand Paris. Nous sommes en train de travailler avec les régions et les métropoles concernées pour trouver le meilleur calendrier,

Madame la ministre, ma question porte sur la réalisation de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur pour relier les trois métropoles régionales Marseille, Toulon et Nice. L'unique ligne ferroviaire existante, créée en 1860, souffre de son ancienneté, avec des problèmes d'infrastructures vieillissantes et des flux tendus permanents, puisque l'ensemble des trains y circulent sans itinéraire alternatif en cas de problème technique. Des noeuds ferroviaires à Marseille ou Nice congestionnent le trafic avec des retards fréquents. Dans les Alpes-Maritimes, la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur est très attendue par les collectivités locales, les opérateurs économiques et les usagers. Elle contribuera à à ouvrir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les autres régions françaises, à désenclaver l'est de ce territoire et à poursuivre la réalisation de l'arc ferroviaire méditerranéen de Barcelone à Gênes. Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures a pris la mesure des problématiques ferroviaires en retenant la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur dans les cinq grands projets prioritaires nationaux. Toutefois, madame la ministre, le rapport précise que les parts respectives des contributions de l'État et des collectivités resteraient similaires à celles actuellement pratiquées, c'est-à-dire des cofinancements proches de la parité pour la plupart des grands projets. Compte tenu de la réforme de la fiscalité locale amorcée avec la suppression de la taxe d'habitation, pouvez-vous garantir aux élus et aux usagers que les décisions que prendra le Gouvernement en matière ferroviaire ne seront pas revues à la baisse en raison d'une réforme ultérieure sur le pacte financier entre l'État et les collectivités

frontalières. Cette mesure pourrait-elle voir le jour dans la loi d'orientation des mobilités et vous semble-t-elle toujours cohérente pour permettre un appui budgétaire supplémentaire aux régions dans le cadre de ces grands projets ferroviaires ?

Pour autant, il ne faudrait pas que la réforme que vous allez engager impose à certains une triple peine. Et c'est bien ce que nombre de territoires, dont celui que je représente, peuvent craindre

... Troisième peine : selon les préconisations d'un rapport qui vous a été remis, ces territoires verraient nombre de leurs lignes secondaires supprimées au mépris de toute logique d'aménagement du territoire et de respect du service dû aux usagers, où qu'ils résident,

les plus peuplés, les plus dynamiques économiquement et aujourd'hui très bien dotés en termes d'infrastructures de transport. Aussi, madame la ministre, j'espère vivement- et je n'en doute pas

peu différente. Le développement des lignes LGV a suscité dans notre pays beaucoup d'espoirs pour le désenclavement des territoires. Pour les liaisons intermétropolitaines et l'accès aux territoires éloignés, voire enclavés, la grande vitesse ferroviaire constitue une alternative pertinente en termes écologiques et économiques aux modes de transport routier et aérien. Le choix du Gouvernement de ralentir, voire de différer ou même d'abandonner, la réalisation d'un certain nombre de grands projets LGV au profit des transports du quotidien peut présenter à court terme une option compréhensible compte tenu des contraintes financières qu'impliquent de tels projets.

dans les dix, quinze ou vingt prochaines années, de compléter le réseau LGV en tenant compte d'impératifs d'aménagement du territoire ? Si le rapport Duron préconise la réalisation à court ou moyen terme, selon les scénarios financiers, des liaisons Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan, il renvoie à beaucoup plus tard l'achèvement de la liaison LGV Rhin-Rhône et la prolongation, à partir de Bordeaux, de la LGV en direction de Dax et de l'Espagne. Par ailleurs la LGV

Si vous réalisiez une carte de France non pas en fonction des distances, mais en fonction des temps de parcours ferroviaire, en prenant Paris et Marseille comme points fixes, Limoges et Clermont-Ferrand seraient au milieu de la Méditerranée et Aurillac proche de la Sicile cette perspective puisse, dans le cadre d'une politique volontariste d'aménagement du territoire, soucieuse de réduire les fractures territoriales et de préserver les chances de développement économique de ces régions, être, à terme, corrigée ?

que je présenterai d'ici à quelques semaines est bien de tenir pleinement compte de ces enjeux d'équité territoriale et d'aménagement du territoire. Nous ne voulons pas laisser de vastes pans de notre pays à l'écart

au mois de juillet dernier, même si le contrat initial qui consistait à mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris n'est pas encore atteint. Lors de cette mise en service, élus et riverains ont constaté que de nombreuses nuisances avaient été sous-estimées. Une

Des mesures sont nécessaires pour vérifier si les concessionnaires ont bien respecté la réglementation acoustique. Il est possible qu'ils

des études en cours. La parole est à M. Michel Savin. Avant toute chose, je tiens à saluer l'intérêt, mais aussi la difficulté, de l'exercice mené par la commission Duron pour cadrer la définition d'une stratégie d'investissement pluriannuelle dans les infrastructures de transport. Toutefois, nombre des conclusions qu'elle présente méritent d'être discutées et critiquées. Certes, d'importants investissements doivent être prioritairement consacrés à l'entretien, à la modernisation et à la régénération des réseaux existants, mais il est essentiel de préserver une part des investissements pour les nouvelles infrastructures qui dynamisent l'économie et préparent l'avenir, dans un contexte de plus en plus concurrentiel avec nos voisins. Il s'agit d'une question de curseur et de volonté politique. À cet égard, les recommandations du rapport Duron concernant les voies d'accès de la liaison Lyon-Turin relèvent du non-sens économique, écologique et géostratégique. Le rapport recommande en effet de repousser les travaux d'aménagement des accès français le Lyon-Turin constitue un ensemble cohérent, qu'il s'agisse des accès ou des tunnels. Cette infrastructure répond à toutes les priorités affichées par votre gouvernement : transition écologique le report modal, compétitivité des entreprises dans les échanges internationaux, relance de la dynamique européenne ... Il s'agit aussi de soutenir la mobilité du quotidien, de Lyon vers les métropoles du sillon alpin. C'est notamment le cas de Grenoble, onzième métropole française avec 450 000 habitants, qui reste, une fois de plus, à l'écart des projets d'aménagement structurants du territoire français. La ligne Lyon-Saint-André-le-Gaz-Grenoble a beau être un point noir connu et reconnu de notre réseau ferroviaire, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers d'usagers, rien n'est fait pour la soutenir. Le report au-delà de 2038 est une entrave forte et durable à la mobilité qui se traduira par un enclavement de la métropole grenobloise. Madame la ministre, le Lyon-Turin est une occasion historique de développer et de moderniser le réseau ferroviaire du sillon alpin. Le Gouvernement

la performance des liaisons TER, des trains de la vie quotidienne, sur les axes Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry, d'autre part. On ne facilite pas la prise de

il paraît raisonnable de réaliser le tunnel de base pour redynamiser ce même trafic et « jouer dans la même cour » que nos voisins, qui ont creusé deux tunnels entre l'Italie et la Suisse et un tunnel entre l'Italie et l'Autriche.

Elle passe par des travaux de régénération de la ligne actuelle Bordeaux-Facture-Dax. Ces travaux doivent être programmés d'ici à 2023 pour améliorer la desserte du sud des Landes, du Pays basque, de Pau et du Béarn.

des délais et à des coûts acceptables à la fois pour les usagers et pour nos partenaires espagnols. Elle seule peut rendre plus ou moins acceptable le report du projet de ligne nouvelle à un horizon postérieur à 2038.

question. Cette ligne a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, ce qui permet de préserver l'avenir et de prendre en compte cette future infrastructure dans les documents d'urbanisme. Par ailleurs, les collectivités des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ont proposé de réfléchir à des ressources financières locales supplémentaires, comme pour la Société du Grand Paris en Nous sommes en train de mener ces travaux avec les collectivités concernées. Nous verrons, compte tenu des ressources disponibles de l'AFITF et des éventuelles ressources complémentaires qui pourraient être dégagées,